En application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique n° 2010 837 et de la loi ordinaire n° 2010 838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission des affaires économiques a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis défavorable par vingt voix contre, et treize voix pour, à la nomination de Mme Emmanuelle Wargon à la présidence du collège de la Commission de régulation de l'énergie. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française

Notre philosophie a été de tendre vers le droit commun, tout en prenant en compte les aspects qui font du territoire polynésien un territoire singulier, atypique, comme beaucoup d'autres, ce qui nous invite à la différenciation. Ce texte, nous l'avons enrichi, ici, au Sénat, sur plusieurs points. Je pense par exemple à l'aménagement des concours

du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

nous sommes parvenus à un texte qui permettra de renforcer l'attractivité de la fonction publique communale en Polynésie française, mais aussi de stabiliser le statut des agents communaux dans leurs rapports avec les mairies et les intercommunalités qui les emploient. Il s'agissait d'abord de faire bénéficier les fonctionnaires des communes de Polynésie française des avancées introduites par les différentes lois relatives à la fonction publique depuis 2011. Qu'il s'agisse des avancées notables en matière d'accès à la fonction publique des communes, de renforcement des droits des fonctionnaires ou encore de modernisation des instances du dialogue social,

et des avancées ont été trouvées jusqu'en commission mixte paritaire, ce qui veut dire que le travail parlementaire, en liaison avec le Gouvernement, s'est exprimé jusqu'au bout. Sur le fond, je me réjouis que l'on tende globalement vers un rapprochement entre le droit commun et les règles polynésiennes, en maintenant des dérogations lorsque les

et qui nous permet de vivre ensemble dans le respect des convictions de chacune et de chacun. Il est précisé que la laïcité, comme l'ensemble des principes déontologiques, s'applique dans les communes de Polynésie sous l'autorité du maire, ce qui est tout à fait normal. Cette précision est utile. J'en viens maintenant aux différents points abordés par M. le ministre et M. le rapporteur. Ce texte comprend des avancées importantes le droit au temps partiel thérapeutique, la possibilité de recruter beaucoup plus facilement des agents reconnus travailleurs handicapés, le télétravail.

Il y a d'abord ce qui relève de l'action sociale. Dans le texte initial, il était prévu que cela pouvait concerner la restauration,

Ensuite, il y a le rétablissement des CAP dans leurs fonctions, c'est-à-dire qu'elles seront nécessairement consultées s'agissant de l'établissement du tableau annuel d'avancement et de la question des mutations, avec les problèmes de changement de résidence que cela pose pour les fonctionnaires. Enfin, je veux évoquer

pas question pour moi de vous faire un laïus sur la Polynésie française et ses spécificités culturelles, humaines et géographiques- chacun les connaît parmi nous. Il n'empêche que, depuis au moins 2017, nous sommes alertés sur le statut des fonctionnaires communaux, inquiets d'être considérés comme une sous-fonction publique. Cette réforme était donc attendue, notamment à la suite des mouvements sociaux qui ont touché l'ensemble des communes. Le Sénat, chambre qui représente les territoires, n'a pas manqué ce rendez-vous, qui devrait permettre la modernisation du régime juridique des plus de 4 700 agents municipaux de Polynésie française

Je tiens donc à saluer le rapporteur pour son travail, ainsi que le regard éclairé de nos collègues polynésiens. C'est un travail important, qui a mis à l'honneur l'esprit du compromis parlementaire et républicain cher au Sénat. Ce compromis s'est traduit par de nombreux apports. Je pense, par exemple, à la possibilité donnée aux communes, à leurs groupements et à leurs établissements de recruter des agents contractuels pour remplacer temporairement les fonctionnaires détachés. Certes, sur d'autres sujets, nous ne sommes pas parvenus à un consensus. Je pense en particulier à l'article 2 relatif à l'accès à la fonction publique des communes par voie d'examen professionnel.

ainsi évoquer l'interdiction des agissements sexistes et du harcèlement sexuel ou la modernisation des règles applicables en matière de déontologie. Mais un sujet a été plus sensible que d'autres sensible que d'autres : la laïcité. L'article 6 qui avait été adopté par notre commission précisait l'obligation de neutralité des fonctionnaires sans se référer à la laïcité.

Une telle disposition serait venue ajouter une crispation regrettable sur un sujet qui fait consensus, à savoir la valorisation du statut des fonctionnaires communaux de la Polynésie française.

la semaine dernière, le Sénat et l'Assemblée nationale se sont accordés sur une rédaction commune, nous permettant d'acter la fin de l'examen parlementaire du projet de loi ratifiant l'ordonnance de 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie

Grâce à cette actualisation, les agents communaux polynésiens bénéficient de nouveaux droits, à l'instar de ceux obtenus par leurs collègues hexagonaux. Aujourd'hui, ils bénéficient d'un congé paternité, d'un congé formation, d'un temps partiel thérapeutique, d'un meilleur encadrement du dialogue social avec leur employeur, d'une protection contre les discriminations liées à une situation familiale ou à une grossesse ou encore d'une protection face aux agissements sexistes et au harcèlement sexuel. Nous mettons les agents à l'abri face aux aléas de la vie et aux comportements répréhensibles, voire condamnables. Par cette ordonnance, la fonction publique est rendue plus moderne et plus attractive recours au télétravail, meilleur dialogue social, adaptations pour des agents reconnus travailleurs handicapés ou encore remplacement de la notation par une appréciation de la valeur professionnelle. Par ailleurs, l'ordonnance prévoit de nouvelles obligations pour nos agents en matière de déontologie et de prévention contre les conflits d'intérêts. Au-delà de ces actualisations,

Ce droit est bien ouvert à tous les contractuels qui se trouvaient en poste au moment du décret de 2005, qu'ils aient ou non explicitement refusé la proposition de reclassement qui leur avait été faite à cette époque. Je vous

ils portent notamment sur la restauration du rôle de contrôle de la commission de déontologie en cas de cumul d'activités ou de départ vers le privé et sur le régime indemnitaire des agents publics. Les autres dispositions restant en discussion ont été soldées lors d'une commission mixte paritaire constructive et bienveillante. Je salue le travail réalisé par ses rapporteurs, Mathieu Darnaud le Sénat et Guillaume Vuilletet pour l'Assemblée nationale. Nous avons notamment pu trouver des solutions en ce qui concerne le respect du principe de laïcité dans nos communes : le maire veillera au contrôle du respect de ce principe déontologique par les agents publics.

le Sénat peut se féliciter d'avoir obtenu la réinscription à l'ordre du jour, après son retrait soudain par le Gouvernement, de ce projet de loi ratifiant l'ordonnance du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction La Haute Assemblée démontre une nouvelle fois son attachement à l'ensemble de nos territoires. L'ordonnance du 8 décembre 2021 est déjà entrée en vigueur. Néanmoins, elle serait frappée de caducité si elle n'était pas ratifiée d'ici à 2023. Il y avait donc urgence à débattre de sa ratification. Prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, cette ordonnance vise à actualiser le statut général des quelque 4 700 agents des communes et des groupements de communes de la Polynésie française. Cette réforme du statut général est très attendue, non seulement par les agents, mais également par les élus. En effet, elle fait suite au vaste mouvement de grève de mai 2017, qui toucha la totalité des communes de la Polynésie française, et résulte d'une longue période de concertation entre les instances locales polynésiennes et le Gouvernement. Prenant en compte les évolutions intervenues dans le droit de la fonction publique communale, l'ordonnance vise à atteindre trois grands objectifs. En premier lieu, elle consolide les droits et les garanties des agents communaux de la fonction publique de la Polynésie française, tout en précisant leurs obligations en matière de déontologie. En second lieu, elle modernise les instances de dialogue social, en confortant le rôle du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française. En dernier lieu, elle améliore l'accès à la fonction publique communale. L'ordonnance vise ainsi à offrir aux agents communaux un cadre juridique clair, stable et protecteur. La commission mixte paritaire a été conclusive ; je ne peux que me réjouir de cet esprit consensuel qui a permis d'aboutir à un texte commun. Toutefois, je voudrais revenir sur un point particulier qui a suscité de nombreux débats : la place très visible qu'occupe la religion dans la vie polynésienne, y compris dans ses dimensions professionnelles et publiques.

l'inscription du principe de laïcité dans le statut général des fonctionnaires communaux ne semblait pas forcément appropriée. Par ailleurs, la loi de 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État n'a jamais été étendue à la Polynésie française.

5 , introduit en séance à l'Assemblée nationale, qui prévoit que le chef de service, agissant sous l'autorité du maire, veille au respect de ce principe. Avant de conclure, je tiens à saluer la qualité des travaux de notre rapporteur, Mathieu Darnaud,

La fonction publique communale de Polynésie française est, comme cela a pu être rappelé au cours des débats précédents, la dernière-née des fonctions publiques de ce territoire, où elle cohabite avec celle de l'État et celle de la collectivité polynésienne.

Éparpillés à travers les cinq archipels du territoire- je pense ici tout particulièrement aux îles Tuamotu -, ces communes et leurs quelque 4 700 agents font en effet face à des contraintes de fonctionnement tout à fait uniques en France.

ordonnance étend aux fonctionnaires communaux polynésiens un certain nombre de droits et de garanties dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux, consolide les outils du dialogue social et ajuste certaines modalités d'accès à cette fonction publique. Lors de l'examen en première lecture de ce texte, notre assemblée avait suivi son rapporteur, Mathieu Darnaud, dont je salue au passage le travail considérable, en complétant cette ordonnance de manière à renforcer la modernisation et l'attractivité de cette fonction publique, mais aussi à mieux l'adapter aux enjeux locaux. Sans revenir dans le détail sur l'ensemble de ces apports, souvent assez techniques, je me bornerai à mentionner l'inscription dans la loi du recours au télétravail, qui est d'une actualité brûlante, la modernisation des procédures de recrutement des personnes atteintes d'un handicap ou encore l'alignement du régime de mise à disposition des fonctionnaires communaux polynésiens sur celui de la fonction publique territoriale.

comme la suppression de la mise à la retraite d'office de la liste des sanctions applicables aux fonctionnaires communaux ou la mise en place d'une voie d'accès à cette fonction publique sur la base d'examens professionnels. Toutefois, les discussions en commission mixte paritaire ont permis d'aboutir à une position d'équilibre avec l'Assemblée nationale, sauvegardant l'essentiel des apports du Sénat et rétablissant plusieurs dispositions précédemment supprimées.

J'avais déjà pu m'exprimer alors sur le symbole très concret que représentait le texte initial du Gouvernement, dans la prise et la ratification d'ordonnances, mais plus encore vis-à-vis des attentes de nos compatriotes polynésiens. Il est toujours bon de rappeler que le précédent a été celui qui a le plus eu recours à des ordonnances ; conjointement, la part d'ordonnances ratifiées est en chute libre, atteignant un taux de 20 % sur le dernier quinquennat, à l'encontre du principe constitutionnel de ratification expresse. Éviter le débat, gouverner seul, encore et toujours : c'était la règle règle des gouvernements de Macron 1 ; nous verrons ce qu'il en est sous Macron 2 ! Cette solitude coupable dans l'exercice du pouvoir est en opposition avec l'équilibre de nos institutions et surtout avec la démarche du Sénat, dont j'espère qu'elle perdurera, car elle est plus nécessaire que jamais dans l'équilibre institutionnel et politique de notre pays. Je tiens à saluer notre collègue Lana Tetuanui pour son engagement en faveur de son territoire et pour les concertations qu'elle n'a cessé de mener, y compris au Sénat, sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Vous le savez, ce territoire compte un peu plus de 4 600 fonctionnaires communaux. Notre rapporteur le rappelait : il était grand temps d'actualiser leur statut. Cette fonction publique communale est une innovation de 2005,

Toutefois, comme l'examen en commission et les auditions menées l'ont montré, cette ordonnance ne correspondait vraiment pas aux demandes locales. D'un point de vue général, la volonté qui s'y faisait jour de se calquer sur le modèle métropolitain

Quant aux questions liées aux finances des communes, si les collectivités en métropole souffrent d'un manque de visibilité sur leurs finances et que l'inaction du Gouvernement sur les problématiques climatiques et ses effets grève leurs budgets,

espérons que celui qui s'ouvre ne lui ressemblera pas trop ! Ce texte reste très fidèle à la vision et à la méthode des derniers gouvernements : une ratification à la carte, des concertations et une prise en compte du terrain insuffisantes, des renoncements inexpliqués.

collègue, mais c'est mon droit de le dire ! Monsieur le ministre, la prise en compte des Polynésiens ne saurait souffrir de ce jeu politique. L'urgence du terrain doit vous obliger, le travail des acteurs de terrain doit vous obliger, la compréhension de l'équilibre de nos institutions doit vous obliger. GEST, pour sa part, prend ses responsabilités ; il votera donc pour ce texte, afin de répondre par des mesures équilibrées aux attentes trop longtemps ignorées de la Polynésie dans la gestion de ses fonctionnaires.

Il aurait été préférable pour nos concitoyens polynésiens qu'il soit voté plus tôt, ce qui aurait montré l'intérêt du Gouvernement pour les collectivités ultramarines et leurs populations. Ce texte nous permet aussi de démontrer l'utilité des luttes sociales.

contre la fonction publique, le gel du point d'indice, le rétablissement de la journée de carence, les suppressions de postes et, plus globalement, la faiblesse de leur pouvoir d'achat. Rappelons que les prix en Polynésie française sont supérieurs de 39 % à ceux de l'Hexagone, selon la dernière enquête de l'Institut de la statistique de la Polynésie française. La vie chère y est donc un défi à relever au quotidien. Ces manifestations ont permis la construction d'un consensus, après des concertations entre les partenaires locaux. Cette fonction publique spécifique à la Polynésie est récente. Pour son évolution et son attractivité, il était nécessaire de lui étendre des dispositions applicables à la fonction publique territoriale. Nous nous félicitons des avancées en matière de lutte contre les discriminations, les agissements sexistes et le harcèlement, mais aussi en matière de déontologie ; à cet égard, je me félicite que notre amendement tendant à attribuer aux fonctionnaires un droit à la consultation d'une commission de déontologie ait été conservé dans la version finale du texte. Ce texte mais réaffirme aussi les devoirs et les valeurs de la fonction publique, qui unit l'ensemble des agents de la République : nous avons défendu le maintien du principe de laïcité, qui a bien sûr vocation à être réapproprié localement, dans le respect de la culture et de l'histoire locales. Nous voterons en faveur de ce texte, car la majorité de ses dispositions bénéficieront aux fonctionnaires communaux polynésiens, mais nous tenons tout de même à émettre des réserves sur certaines mesures. Malheureusement, en toile de fond de ce texte, nous retrouvons la logique de la loi de transformation de la fonction publique et ses dogmes libéraux : l'encouragement à la contractualisation, le rétrécissement du champ d'action des instances représentatives du personnel ou encore le remplacement de la notation par un entretien individuel d'appréciation de la valeur professionnelle. Tout cela va, selon nous, vers une casse du statut et une précarisation des agents. Nous aurions également aimé que le texte aille plus loin dans la reprise des propositions du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, par exemple en adoptant

ne pourront évidemment être atteintes si l'on ne s'en donne pas les moyens. Il est insupportable que ces agents qui défendent l'intérêt général au quotidien ressentent une mise à l'écart statutaire ; un tel texte contribue à y remédier. Mais les communes polynésiennes subissent de fortes contraintes budgétaires et l'État doit mieux les accompagner financièrement. C'est une nécessité, pour améliorer l'évolution professionnelle des agents et pour atteindre les objectifs de politiques publiques défendus dans un tel texte, comme l'action sociale. Le rapport demandé au Gouvernement à l'article 23 sera donc le bienvenu pour mettre en lumière ces besoins. Vous le savez, monsieur le ministre, nous sommes opposés à la pratique des ordonnances, lorsqu'elles sont utilisées pour légiférer sur les collectivités ultramarines. Toutefois, nous voterons ce texte important pour nos concitoyens polynésiens, un texte qui a pu susciter un consensus entre les acteurs concernés, malgré les points de vigilance que nous avons soulevés. Je tiens pour finir à saluer particulièrement notre collègue Lana Tetuanui,

Tout vient à point à qui sait attendre et il n'est jamais trop tard pour bien faire, me dira-t-on ! Aussi, sans refaire l'histoire, je rappellerai néanmoins que la fonction publique consacrée aux seules communes de Polynésie française est récente : elle n'est effective que depuis l'ordonnance de 2005, actualisée en 2011, et comprend à ce jour 4 935 agents, dont 1 316 contractuels. Or il aura fallu un large mouvement de contestation, en 2017, pour que le gouvernement central se penche sérieusement sur le sujet, afin de répondre aux quelques revendications de nos agents communaux, qui manquaient de certains droits, et non des moindres. L'objectif de ce projet de loi est de rendre plus attractive la fonction publique communale et d'inciter notre jeunesse polynésienne à s'inscrire aux concours pour servir nos 48 communes et 98 communes associées. peuvent parfois paraître excessifs, mais notre spécificité bien particulière à l'égard de toutes les autres collectivités ultramarines, c'est bien notre configuration géographique,

Évitons de copier et coller le modèle métropolitain, inadapté à nos structures locales ! Néanmoins, je me réjouis des avancées obtenues sur des sujets parfois très techniques et je tiens à saluer le travail remarquable des rapporteurs,

le Parlement a complété l'ordonnance par le report du droit d'option jusqu'en décembre 2023 ; l'institution d'une plus grande souplesse dans les conditions de remplacement des agents et dans le dispositif de mise à disposition le maintien des compétences des CAP ; la réintroduction des missions des CTP ; l'adaptation du droit de la déontologie et le maintien de la commission locale instituée en 2005 ; l'adaptation de l'action sociale conformément aux attributions dévolues à nos communes la correction de l'article 38 de l'ordonnance sur le recrutement ou le reclassement des catégories C et D ; l'aménagement des conditions et des modalités des concours des travailleurs handicapés le placement sous l'autorité du maire du respect du principe de la laïcité, auquel M. Sueur s'était montré très attaché ; le maintien de la réserve opérationnelle avec saisine du Conseil supérieur de la fonction publique

votre rappel du respect du principe de la libre administration de nos communes. Toutes ces évolutions vont dans le bon sens et je me félicite du travail laborieux qui a été accompli. Pour conclure,

pour nos outre-mer. Le groupe Union Centriste votera ce projet de loi ; je vous en remercie.

La séance est suspendue. La séance est reprise. L'ordre du jour appelle une déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, en application de l'article 50-1 de la Constitution, sur le projet de programme de stabilité pour 2022-2027.

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, en application de l'article 50-1 de la Constitution, j'ai l'honneur de vous présenter le programme de stabilité pour la période 2022-2027, qui sera prochainement transmis à la Commission européenne. Comme chaque année, ce programme détaille les prévisions de croissance et la trajectoire de finances publiques que le Gouvernement a déterminées. Mais je veux dire d'emblée que ce programme de stabilité est aussi l'occasion de réaffirmer ce qui est le coeur de notre stratégie en matière d'économie et de finances publiques. Ce programme de stabilité est avant tout un programme dédié à la croissance et au plein emploi. En 2017, le Président de la République s'était engagé à sortir notre pays du chômage de masse.

Nous l'avons fait grâce à nos réformes, en particulier la réforme du marché du travail, engagée dès l'été 2017 pour redonner aux employeurs des capacités à embaucher et à créer des emplois dans notre pays. De fait, nous avons créé près de 1,3 million d'emplois en cinq ans : ce sont 1,3 million de Français qui ont retrouvé un travail, un espoir et une dignité parce que notre majorité a su mener ces réformes. la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a révolutionné l'accès à l'apprentissage et à la formation : il y a cinq ans, notre pays comptait moins de 300 000 nouveaux apprentis chaque année ; il en compte aujourd'hui plus de 700 000. C'est une formidable réussite pour l'insertion de nos jeunes dans la vie active et une formidable victoire contre le chômage. Aujourd'hui, ce qui paraissait impossible est à portée de main : oui, le plein emploi est possible dans notre pays ! Il sera atteint, parce que nous allons poursuivre les réformes et lever tous les freins à l'accès à l'emploi.

Dans l'industrie, les déclarations d'embauche progressent de 9,6 % sur un an. C'est une victoire pour l'emploi, mais aussi pour le financement de notre protection sociale, puisque la masse salariale soumise à cotisations a progressé de 11 % en un an et dépasse désormais de 7,7 % son niveau d'avant-crise. Alors, nous allons poursuivre et accentuer nos efforts pour atteindre le plein emploi d'ici à 2027 autour de trois grands axes. Ce sera, tout d'abord, la réforme de France Travail, pour mettre davantage en réseau les services de Pôle emploi et les services des collectivités dédiés à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et notamment des allocataires du Depuis un an, le nombre de foyers touchant le RSA recommence à baisser, parce que nous créons des emplois, mais il nous faut aller plus loin. Comme le Président de la République s'y est engagé, nous renforcerons leur accompagnement et l'effort de la collectivité pour permettre leur véritable insertion dans l'emploi.

la réforme de l'assurance chômage vise à assurer que chaque Français trouve toujours un gain au travail et à faire en sorte que celui-ci soit mieux rémunéré. Je rappelle qu'avec ses hausses successives, y compris celle qui est intervenue voilà quelques jours à hauteur de 2,01 %, le SMIC a augmenté de 8 % sur un an.

cependant continuer à assurer ce gain au travail ; Olivier Dussopt mènera dès la rentrée prochaine une concertation en ce sens avec les partenaires sociaux pour modifier de nouveau les règles de l'assurance chômage. est l'objectif numéro un de ce programme de stabilité : favoriser la croissance pour atteindre le plein emploi. Je viens d'exposer les réformes que nous engageons pour y parvenir. Ce programme de stabilité traduit un autre engagement fondamental pris par le Président de la République durant la campagne présidentielle celui de tenir nos comptes. Avant de présenter le cadre général, permettez-moi de revenir sur le contexte économique dans lequel nous sommes. Vous le savez, la très forte reprise économique en 2021 après la levée des restrictions imposées par l'épidémie de covid-19 et l'invasion de l'Ukraine depuis le mois de février dernier nous ont fait entrer dans une période de forte hausse des prix. Cette dynamique, nous l'avions anticipée, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons pris des mesures dès l'automne dernier et inscrit deux textes à l'ordre du jour de cette session extraordinaire, contenant plus de 20 milliards d'euros de mesures supplémentaires pour protéger nos compatriotes. Les choix que nous faisons, les mesures que vous défendez et adoptez dans cet hémicycle ont un impact direct sur l'évolution de l'inflation. Je rappelle d'ailleurs que l'Insee a estimé que les mesures du « bouclier tarifaire » sur le gaz et l'électricité prises dès l'automne dernier ont permis d'éviter 2 points d'inflation à nos compatriotes. Cette dynamique de stabilisation de l'inflation est désormais enclenchée. Je rappelle les prévisions qui ont été relayées par Bruno Le Maire : l'inflation qui atteindrait son pic dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois commencerait à décroître pour réellement baisser dans le courant ou à la fin de l'année 2023. Nous restons évidemment tributaires de l'évolution des marchés mondiaux et du contexte géopolitique. que cette probable stabilisation nous permet, dans le cadre de ce programme de stabilité, de tabler sur un atterrissage à 5 % en moyenne cette année, suivi d'une hausse de 3,2 % en 2023, avant de redescendre sous la barre des 2 % au courant de l'année 2024, en cohérence avec l'objectif de la Banque centrale européenne. Autre bonne nouvelle que je veux partager avec vous : le chiffre de la croissance de 0,5 % pour le deuxième trimestre. Ce signal positif atteste du dynamisme et de la robustesse de notre économie, malgré le climat d'incertitude qui pèse notamment sur la consommation des ménages. Concrètement, cela veut dire que nous avons d'ores et déjà acquis 2,5 % de croissance cette année, conformément à l'objectif révisé que nous avons fixé. Est-ce à dire que nous avons conjuré toutes les menaces ou relevé tous les défis ? Évidemment non, mais, dans cette période où l'inquiétude gagne les ménages comme les entreprises, il me semble essentiel de rappeler qu'il existe un scénario favorable : celui de la croissance, du plein emploi, de la maîtrise des prix et de la tenue de nos comptes. les sénateurs, voilà la situation dans laquelle nous sommes. La transmission de ce programme de stabilité intervient donc à un moment charnière, puisqu'il marque l'avènement d'une phase de normalisation pour nos finances publiques. Oui, c'est un programme de normalisation après la parenthèse du « quoi qu'il en coûte », durant laquelle nous avons mis en place les amortisseurs indispensables face à la pandémie la plus grave depuis un siècle. Nous sommes passés du « quoi qu'il en coûte » au « combien ça coûte ».

Je rappelle d'ailleurs que la charge de la dette a bondi de 17 milliards d'euros en comptabilité nationale cette année, principalement du fait de l'inflation et de la remontée des taux. Je sais que, sur certaines travées, les mots « analystes », « investisseurs », « agences de notation » peuvent susciter une forme de rejet ou de circonspection. Oui, certains d'entre vous admettent difficilement que la sixième puissance mondiale doive intégrer la contrainte des taux d'intérêt et la pression qu'elle exerce. À ceux-là, je répondrai, d'une d'une part, que tout État, aussi puissant soit-il, doit composer avec cette réalité dès lors qu'il est confronté à un besoin de financement structurel, d'autre part, que la bonne manière d'appréhender le sujet, ce n'est pas d'entretenir le mythe du non-remboursement, c'est de faire le choix de tenir nos comptes. Il n'y a ni indépendance ni capacité d'action sans des finances maîtrisées. maîtrisées. Celles et ceux qui défendent la souveraineté devraient donc soutenir la trajectoire responsable que nous présentons aujourd'hui. Oui, ce programme de stabilité traduit d'abord l'objectif qui est le nôtre en matière de maîtrise des comptes publics. Le chemin que nous empruntons doit nous permettre de ramener le déficit public sous le seuil de 3 % à l'horizon 2027. Corrélativement, le poids de la dette publique dans le PIB commencerait à décroître à compter de 2026. Je l'ai indiqué au début de mon propos : ce programme n'est pas seulement une feuille de route pour nos finances publiques, c'est le cadre macroéconomique dans lequel nous allons évoluer et qui doit nous permettre d'atteindre nos objectifs. Ceux-ci sont clairs : protéger les Français face à la hausse des prix de l'énergie, tout en menant des réformes d'ampleur pour soutenir la croissance, accélérer la transition écologique et atteindre le plein emploi.

intègre logiquement les mesures annoncées par le Président de la République au cours de la campagne électorale. Je pense aux mesures en faveur du pouvoir d'achat des Français, dont nous avons débattu encore longuement cette nuit, et de la compétitivité des entreprises

La soutenabilité des finances publiques ne doit pas se faire par le biais d'efforts supplémentaires demandés par l'impôt aux Français. Dans les cinq prochaines années, il n'y aura pas de hausse généralisée des prélèvements obligatoires.

Je rappelle que le programme de stabilité intègre une hausse de la dépense publique de 0,6 % en volume sur la période 2023-2027. C'est, je le souligne, l'augmentation de la dépense publique la plus faible depuis vingt ans, ce qui atteste de notre détermination à tenir nos comptes. À celles et ceux qui dénoncent un agenda caché fait de coupes brutales et de réductions massives d'effectifs, j'oppose le démenti le plus catégorique : nous ne réduisons pas la dépense, nous gérons le rythme de son augmentation. Magnifique ! En clair, nous faisons en sorte que la dépense publique augmente moins vite que la richesse que nous créons. Pour tenir l'objectif d'augmentation annuelle de la dépense publique de 0,6 % en moyenne, il faut que l'effort soit réparti entre l'État, les collectivités territoriales et la sécurité sociale. Concrètement, cela doit se traduire par une baisse en volume de 0,4 % sur la norme de dépenses pilotables de l'État et de 0,5 % sur les dépenses de fonctionnement des collectivités locales. durant cette période, nous faisons le choix suivant : si la norme des dépenses de l'État baisse en volume et si les dépenses de fonctionnement des collectivités locales doivent aussi être maîtrisées en volume,

Le Gouvernement aura l'occasion d'exposer de manière détaillée l'ensemble des mesures mises en oeuvre pour assurer cette stratégie, lors de la présentation du projet de loi de programmation des finances publiques, à la rentrée prochaine. viens à la croissance. J'ai déjà dit un mot de la bonne nouvelle s'agissant des chiffres du deuxième trimestre et de notre capacité à atteindre l'objectif de 2,5 % fixé pour cette année. Par la suite, la croissance serait de 1,4 % en 2023, puis accélérerait sur la période 2024-2027, passant de 1,6 % à 1,8 % entre 2024 et 2027. En 2023, le rebond serait ralenti par la situation géopolitique et les tensions en matière d'offre, mais resterait soutenu par les mesures de soutien au pouvoir d'achat. Il serait plus marqué à partir de 2024 et s'accélérerait jusqu'en 2027, pour s'établir à 1,7 % en moyenne sur la période 2024-2027.

Il s'agit d'une hausse de 15 points par rapport à 2019, mais d'une baisse de plus de 2 points par rapport à 2020. En 2022, le ratio d'endettement devrait baisser légèrement, malgré les mesures visant à protéger les Français du contexte inflationniste, du fait notamment de la poursuite de la croissance, et atteindrait 111,9 %.

Nous avons réduit le déficit public de 2,5 points de PIB l'année dernière et nous tiendrons la cible de 5 % cette année, inchangée depuis la loi de finances initiale votée à l'automne dernier. D'abord, la croissance est conforme à nos prévisions, comme l'a confirmé l'Insee voilà quelques jours. Ensuite, l'impact budgétaire des mesures que nous avons mises en place pour soutenir le pouvoir d'achat est en grande partie compensé par les économies réalisées sur les charges de service public de l'énergie. Enfin, nous pouvons compter sur un surplus de recettes fiscales lié à l'exceptionnel rebond de l'économie française l'année dernière. Sur la période 2023-2027, le Gouvernement s'est fixé pour objectif le retour à des comptes publics maîtrisés- c'est la normalisation que j'évoquais au début de mon propos. Le déficit public devrait revenir sous le seuil de 3 % à l'horizon 2027, grâce à un ajustement structurel de 0,3 point de PIB par an à compter de 2024. Cela doit conduire à une décrue du ratio dette publique/PIB à compter de 2026. Cette maîtrise des finances publiques ne fait en aucun cas obstacle aux investissements indispensables pour assurer la transition écologique et numérique, atteindre le plein emploi et s'assurer de la compétitivité de nos entreprises- j'ai déjà évoqué la suppression à venir de la CVAE. Cette trajectoire s'inscrit en cohérence avec les plans France Relance et France 2030, qui permettront de soutenir l'activité et le potentiel de croissance, en accélérant la transition écologique, en favorisant l'investissement, l'innovation, la cohésion sociale et territoriale et en assurant la souveraineté numérique et industrielle.

nous nous retrouvons aujourd'hui pour débattre du programme de stabilité que le Gouvernement s'apprête à transmettre aux institutions européennes et qui décrit le scénario macroéconomique et la trajectoire des finances publiques pour les années 2022 à 2027.

puis « début juin », puis « après les élections législatives », puis « début juillet ». Enfin, début août, nous y sommes : il est là. Pourquoi un tel retard ? Pourquoi avoir eu besoin de trois mois supplémentaires pour présenter ce programme de stabilité ? Certains pensent que le Gouvernement aurait pu vouloir cacher aux électeurs, le temps de la campagne des législatives, ses véritables ambitions et son programme pour le redressement des finances publiques. Toutefois, pour que cette hypothèse tienne, il aurait fallu que le programme de stabilité témoigne d'une ambition et comporte un programme pour la consolidation des finances publiques. Or, dans ce document, vous ne trouverez ni l'un ni l'autre, Pour commencer, le programme de stabilité retrace un scénario macroéconomique qui me paraît pour le moins optimiste. La prévision de croissance du PIB en volume pour l'année 2022 est de 2,5 Je me réjouis, sur ce point, des bonnes nouvelles annoncées par l'Insee la semaine dernière indiquant que l'activité avait augmenté de 0,5 % au deuxième trimestre 2022, alors qu'elle s'était contractée au premier trimestre.

Pour les années 2024 à 2027, j'ai aussi le sentiment que le scénario de croissance du PIB est, à ce stade, très au-dessus de ce que nous pouvons sérieusement attendre. Imaginez : d'après les prévisions du Gouvernement, le PIB devrait augmenter en volume de 12,6 % entre 2021 et 2027, alors que, dans le scénario du FMI, l'on atteindrait seulement 9,4 %. Cet écart représente- excusez du peu ! -45 milliards Il est probable que cette surévaluation de la croissance économique soit liée partiellement à une prévision trop optimiste quant à l'évolution du taux de chômage, avec seulement 5,2 % en 2027 d'après les données du programme de stabilité, contre 7,4 % selon le FMI. Les hypothèses du programme de stabilité concernant l'écart de production me paraissent décalées par rapport à la réalité de notre économie. En effet, le Gouvernement estime que notre économie évoluera, au moins jusqu'en 2023, de près d'un point de pourcentage en dessous de son niveau potentiel.

C'est ensuite une hypothèse qui permet d'anticiper des taux de croissance plus forts, puisqu'un écart de production négatif et important signale que l'économie bénéficie d'un fort potentiel de rebond. C'est enfin une hypothèse qui n'est partagée que par l'OFCE. Ainsi, la Commission européenne estime qu'en 2023 l'économie évoluera déjà à son niveau potentiel. par le programme de stabilité quasiment tout au long de la période 2022-2027 s'expliquerait non seulement par l'hypothèse d'un écart de production négatif très important en 2022, mais surtout par une prévision de croissance potentielle de 1,35 qui me paraît surestimée. J'observe que, d'après le Gouvernement, la croissance potentielle serait principalement soutenue par certaines réformes du marché du travail et de l'emploi : réforme des retraites et de l'assurance chômage, par exemple. Or, pour l'essentiel,

Pourtant, comme l'a très justement relevé le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), ces hypothèses sont très optimistes si l'on tient compte du fait que la demande de biens et services de nos partenaires pourrait progresser moins rapidement qu'anticipé et que le resserrement de la politique monétaire et des conditions de financement devraient, au contraire, ralentir la progression des investissements. Le scénario macroéconomique du programme de stabilité repose donc sur des hypothèses que je juge précaires et peu détaillées. En tout état de cause, c'est sur ce scénario macroéconomique qu'est construite la trajectoire des finances publiques retenue par le Gouvernement.

soit une augmentation, hors mesures de soutien face à la crise sanitaire et à l'inflation, de plus de 250 milliards d'euros par rapport à 2022. On peut relever que le Gouvernement s'engage à ne laisser progresser les dépenses publiques en volume que de 0,6 % par an en moyenne. En pratique, cet effort ne concernera que les seules années 2024 à 2027, puisque les dépenses publiques neutralisées des mesures de soutien face à la crise sanitaire et à l'inflation progresseront de 3,5 Ainsi, rapporté à l'ensemble du quinquennat, l'effort consenti consistera en une croissance moyenne en volume des dépenses publiques ordinaires de l'ordre de 1,2 % par an et non de 0,6 %. On peut également observer que le Gouvernement propose de faire peser les efforts sur la seconde moitié du quinquennat plutôt que sur le début, ce qui ne manque pas de surprendre. Chacun sait en effet que c'est en début du quinquennat que les mesures les plus volontaires, éventuellement les plus difficiles à prendre, doivent être décidées. Finalement, avec un effort aussi limité, notre déficit public refluera assez lentement et ne reviendrait en dessous de 3 % du PIB qu'en 2027, et encore de 0,1 point Notre endettement public continuerait de s'accroître et ne refluerait qu'en 2027 pour revenir au même niveau que l'année dernière, c'est-à-dire 112,5 % du PIB. cette trajectoire manque aussi de réalisme : aucune documentation ne l'accompagne. Ainsi, d'après ses propres estimations, la trajectoire de dépense du Gouvernement représenterait une économie d'environ 45 milliards d'euros en 2027 par rapport à un scénario à législation inchangée. Au-delà de la réforme des retraites régulièrement mise en avant par le Gouvernement, alors qu'elle ne produira pas d'effets budgétaires à court terme, je relève qu'une bonne part des économies attendues pourrait

stade, revendiquer un objectif global d'économies des dépenses publiques dont la réalisation repose sur des perspectives d'évolution du marché de l'emploi aussi fragiles que celles qu'a retenues le Gouvernement ne me paraît pas sérieux. Mes chers collègues, je prends acte aujourd'hui du fait que le Gouvernement s'est contenté du service minimum pour construire ce programme de stabilité, en retenant des hypothèses macroéconomiques et de maîtrise des dépenses que j'estime peu crédibles. J'espère très sincèrement que, comme l'y a invité le Haut Conseil des finances publiques, le Gouvernement fera preuve de plus de sérieux dans la préparation du projet de loi de programmation des finances publiques, que nous attendons Ce texte devra notamment décrire les moyens que le Gouvernement entend mobiliser pour réduire la dépense de l'État de 0,4 % en volume et celle des collectivités locales de 0,5 % en volume, en moyenne, jusqu'à la fin du quinquennat. J'espère tout aussi sincèrement que les engagements de maîtrise des dépenses qui y figureront seront plus ambitieux, mais surtout plus crédibles et mieux documentés que ceux qui figurent aujourd'hui dans ce programme de stabilité. Alors même que nous assistons à un changement de régime dans le financement de notre endettement public, nous avons l'obligation de démontrer notre sérieux en matière budgétaire. Pour conclure, je rappelle que toutes les économies que les administrations publiques sauront dégager sont autant de ressources que nous pourrons mobiliser pour engager la réduction de la dette écologique, qui préoccupe à juste titre les jeunes générations et, à vrai dire, tous les Français. C'est assurément un défi que nous devons relever ensemble. La parole

Il y a peu, certains étaient diabolisés en raison de leur supposée désobéissance aux règles européennes ; aujourd'hui, surprise, ce sont ceux-là mêmes qui se présentaient comme les hérauts de la européenne qui se permettent de désobéir à ces règles

sortants. Circonstance aggravante, nous nous retrouvons pour en débattre au début du mois d'août, dont on conviendra qu'il s'agit d'une période particulièrement peu favorable à un débat parlementaire approfondi. Comme pour les autres textes de finances publiques, monsieur le ministre, vous avez fait le choix de retarder le calendrier à l'extrême, ce qui n'est absolument pas satisfaisant. Quelques indiscrétions concordantes, rapportées par la presse, nous indiquent cependant que vous auriez demandé à votre administration de tordre quelque peu les chiffres pour que ceux-ci soient raccord avec votre discours. Ceci explique peut-être cela Que dire, qui plus est, du fait que l'information est transmise à la presse plus de dix jours avant de l'être au Parlement, mettant celui-ci dans l'impossibilité de répondre aux affirmations souvent péremptoires du Gouvernement ? C'est une méthode absolument inadmissible Ce point étant rappelé, je tiens à dire combien ce document peut laisser perplexe, comme d'ailleurs cela transparaît dans l'avis très réservé du Haut Conseil des finances publiques. Bien sûr, nous avons l'habitude, comme la Commission européenne malheureusement, que le programme de stabilité français soit optimiste, peu crédible, renvoyant régulièrement les mesures les plus difficiles pour la fin de la période- prière d'y croire

Cependant, la leçon devrait nous servir : l'ampleur des incertitudes géopolitiques et macroéconomiques doit, me semble-t-il, nous inciter à davantage de prudence, à tout le moins, à présenter des scénarios plus étayés. Je ne reviens pas sur les chiffres fournis tout à l'heure par le rapporteur général, mais je ne peux que souligner l'existence d'aléas très négatifs, comme les qualifie le HCFP : baisse de la croissance en Allemagne, conflit en Ukraine, difficultés de la Chine, etc. Je doute aussi Je doute aussi que votre scénario intègre l'effet récessif des mesures de ralentissement de la dépense publique que vous préconisez par ailleurs, monsieur le ministre. Selon vos termes, vous prévoyez l'augmentation en volume de la dépense publique la plus faible depuis vingt ans. En raison du contexte politique et social, cela ne semble ni raisonnable ni réaliste,

Pour les administrations publiques locales, les modalités de leur contribution sont pour le moins nébuleuses. Les administrations de sécurité sociale devront participer à l'effort avec la poursuite de la transformation du système de santé, dont on ne mesure pas bien les effets en termes d'économies.

Concernant les recettes, vous annoncez une poursuite des baisses d'impôts, tournées cette fois vers les seules entreprises, au nom d'une « politique de l'offre » qui viendra fragiliser encore davantage nos finances publiques. Je doute fort que le problème de compétitivité de nos entreprises relève avant tout d'un problème fiscal. vous évoquez la remise en cause de niches fiscales et sociales peu efficaces, mais sans aucune illustration ni chiffrage. Bref, vous ne dites rien ! Quoi qu'il en soit, il me semble plus que jamais nécessaire de consolider nos recettes fiscales pour financer les politiques publiques dont notre pays a besoin, notamment en matière d'investissements. J'espère que le projet de loi de programmation des finances publiques précisera une trajectoire des finances publiques aujourd'hui à peine ébauchée et, au fond, peu crédible en l'état. Finalement, monsieur le ministre, votre feuille de route budgétaire ressemble franchement plus à une mise en garde pour vos collègues dépensiers du Gouvernement qu'à une proposition sérieuse transmise à la Commission européenne et aux parlementaires. La parole

des dépenses publiques. Ce programme souligne ce que la commission des affaires sociales a déjà pu observer par elle-même : après un exercice 2020 extraordinaire à tous égards, les dépenses de la sécurité sociale, à commencer par celles de la branche maladie, ont encore crû fortement en 2021. La hausse restera significative en 2022. Seul un bond spectaculaire des recettes, principalement sous l'effet de l'évolution de la masse salariale, a permis de contenir quelque peu les déficits, à un niveau cependant très élevé : 24 milliards d'euros en 2021. En revanche, je me réjouis de l'amélioration de la situation financière de l'assurance chômage, en espérant qu'elle sera durable et qu'elle permettra au régime de retrouver un niveau d'endettement supportable. Pour l'avenir, de façon assez traditionnelle, le programme de stabilité dessine une trajectoire financière optimiste, qui demande à être vérifiée, notamment pour ce qui concerne l'accélération de la croissance, que vous anticipez à partir de 2024. De ce fait, prises dans leur ensemble, les administrations de sécurité sociale retrouveraient une capacité de financement dès 2022, leur excédent global atteignant même 1,3 % du PIB en fin de période. J'en prends acte. Néanmoins, je tiens à souligner que les dernières lois de financement de la sécurité sociale dessinaient une trajectoire financière bien plus sombre, incompatible avec l'extinction de la dette de la sécurité sociale avant la fin de l'année 2033, comme l'impose d'ailleurs la loi organique en vigueur.

Tout juste est-il précisé que « la maîtrise des dépenses publiques repose principalement sur des réformes structurelles, la réforme des retraites Vous indiquez ensuite que « le Gouvernement aura l'occasion d'exposer de manière détaillée l'ensemble des mesures mises en oeuvre pour assurer cette stratégie à l'automne, lors de l'élaboration de la nouvelle loi de programmation des finances publiques ». Nous continuerons donc d'attendre.

Mon dernier mot sera pour souligner que le programme de stabilité revient assez longuement sur les évolutions du cadre organique des lois de finances. Le Gouvernement y voit un outil qui permettra au Parlement de mieux contrôler les finances publiques. Je me permettrai simplement de vous rappeler, monsieur le ministre, que le cadre organique des lois de financement de la sécurité sociale changera, lui aussi, dès le mois de septembre, grâce à l'entrée en vigueur de la loi organique du 14 mars 2022. Bien que ce texte n'ait pas repris les propositions les plus ambitieuses du Sénat, il devrait permettre, si nous le faisons vivre, d'améliorer le contrôle parlementaire sur les finances sociales, notamment grâce à une disposition importante : la clause de retour au Parlement en cas de dérapage en cours d'exercice. Il reviendra à chacun d'entre nous de nous emparer de ces outils. Pour sa part, monsieur le ministre, le Gouvernement devra se départir de l'idée solidement ancrée, comme nous l'avons encore vérifié en 2020 et en 2021,

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, de programme de stabilité nous est présenté avec plusieurs mois de retard, cela a été dit, et nous est transmis dans un délai qui frise l'irrespect du Parlement. Même si rien ne vous oblige, quel mauvais signal en ce début de mandature ! Nous y étions habitués sous le précédent quinquennat, mais nous avions un peu d'espoir, puisque nous pensions avoir compris que le Gouvernement voulait favoriser le dialogue avec les parlementaires. M. le ministre nous disait il y a encore une semaine combien il était important de laisser le Parlement travailler en amont sur les textes. Visiblement, cela reste pour l'instant un voeu pieux Sur le fond, ce document soulève des interrogations en raison notamment de l'insuffisance des informations fournies. Ainsi, on comprend que la stratégie gouvernementale se fonde sur une réduction de la dette à compter de 2026 et sur un passage sous la barre des 3 % du déficit en 2027.

Au regard du contexte économique et social, d'une part, et de la dynamique naturelle de la dépense publique, d'autre part, comment allez-vous vous y prendre ? Nous sommes en droit de partager l'analyse du Haut Conseil des finances publiques, qui parle d'une trajectoire de finances publiques qui s'appuie sur une prévision de croissance un peu trop optimiste, sur des réductions de dépenses à ce stade non documentées par une description précise des réformes et des mesures en dépenses. J'évoquerai tout d'abord vos prévisions de croissance trop optimistes.

des impôts de production, des réformes des retraites, du marché du travail, de la formation, du chômage, du RSA, mais aussi de la poursuite des dépenses des plans France Relance et France 2030. Mais la réalité sera tout autre, monsieur le ministre ! La cure d'austérité que vous allez imposer aux Français du fait de la baisse continue des dépenses publiques en valeur réelle, notamment pour le financement des services publics, et de l'insuffisance des revalorisations des dispositifs sociaux,

Pourtant, nous savons qu'une hausse des dépenses en volume est prévue pour financer le Ségur de la santé, le plan d'urgence pour l'hôpital public et le plan urgences. Pourquoi ne disposons-nous pas de chiffres précis ? du financement du cinquième risque, qui a aujourd'hui totalement disparu des radars et dont on connaît pourtant l'impact budgétaire ?

souvent pour compenser le retrait de l'État dans les territoires, et, d'autre part, qu'elles réalisent 70 % des investissements publics. Vous prévoyez qu'elles seront de nouveau associées à l'effort de maîtrise de la dépense publique. Attention à ne rien briser briser ! Vous vantez dans ce document les bons résultats obtenus en matière de baisse du chômage. Vous avez un art certain d'enjoliver la réalité ! Il faut mettre cette baisse en relation avec une augmentation des dispositifs conduisant à une sortie du chômage, notamment les contrats en alternance et les contrats d'apprentissage.

D'une manière générale, vous ne pouvez pas évacuer la question de l'explosion de la paupérisation de nos concitoyens. La crise sanitaire a augmenté d'un million le nombre de pauvres dans notre pays ; ceux-ci représentent désormais 14,6 % de la population. Cela explique, selon le rapport du Secours catholique, que 7 millions de Français aient eu recours à l'aide alimentaire en 2021. À l'autre bout de la chaîne, au contraire, une petite élite peut s'estimer très satisfaite de votre politique, car c'est pour elle que vous gouvernez depuis maintenant cinq ans. En cinq années, Emmanuel Macron a ainsi supprimé 80 milliards d'euros de recettes fiscales pérennes. Les commentateurs économiques insistent beaucoup sur le « quoi qu'il en coûte » des dépenses du Président. Il ne faudra pas oublier désormais d'y ajouter le « quoi qu'on en perde » des recettes

Si la crise sanitaire a fait exploser les budgets et gonfler la dette, le cap demeure le même : pas de contreparties aux aides de l'État, pas de mise à contribution des très riches à l'effort national. Pis, malgré le Ségur, on continue de fermer des lits d'hôpital, car le paradigme gestionnaire à courte vue perdure. De même, la crise sanitaire mondiale, la guerre en Ukraine, les tensions sur les prix de l'énergie, l'inflation qui croît, tout ce cocktail a révélé la nécessité d'un changement de politique de grande envergure. Nous n'avons plus le choix : nous devons désormais nous prémunir contre les crises à venir et protéger les plus vulnérables d'entre nous. Il nous faudra atténuer, voire résoudre, les crises, qu'elles soient sociales, économiques ou écologiques, et résorber les inégalités qui fragilisent la cohésion sociale et la démocratie. Il n'est plus tenable de faire « en même temps » des cadeaux fiscaux aux plus riches et de prétendre vouloir soutenir les plus démunis avec des primes ou des baisses éphémères de quelques centimes des prix à la pompe. Le ruissellement ne fonctionne pas et la loi du marché ne réduit pas les inégalités.

rétorquera volontiers qu'il serait également bon que le Gouvernement cesse de penser que, face à chaque défi, la solution consiste à baisser les impôts ! Un État fort est un État capable d'agir, grâce à des marges budgétaires importantes issues des recettes fiscales.

pour accroître notre souveraineté économique. Sauf à tuer nos services publics et à décourager définitivement ceux qui voudraient y travailler- je pense aux soignants et aux enseignants -, il faudra bien améliorer les conditions de travail et de rémunération.

an. D'autres solutions existent. À l'échelon européen, il nous faut déjà redéfinir un cadre budgétaire et monétaire durable et rebâtir nos politiques à la hauteur des enjeux qui sont devant nous. À cet égard, une question devient de plus en plus prégnante, celle des ressources propres. L'adoption de la taxe de 15 % sur les multinationales est actuellement bloquée par un veto hongrois,

D'autres ressources peuvent être mobilisées : le scandale des, qui a révélé que 11 300 milliards de dollars étaient placés dans des paradis fiscaux, nous rappelle l'urgence pour les États membres de coopérer entre eux afin de renforcer la transparence et, ainsi, de mettre un terme à ces pratiques fiscales dommageables. Un système fiscal plus équitable à l'échelle européenne est un impératif pour mieux lutter contre les inégalités en matière de revenus et de richesse. Il devient essentiel de franchir le pas vers une fiscalité commune. Il est désormais temps de mettre en place une imposition commune des bénéfices bénéfices des sociétés et de conclure les négociations afin d'instaurer une taxe sur les transactions financières d'ici à 2026. Enfin, nous devons revenir sur ces règles budgétaires européennes-

Leur suspension pendant la période de pandémie est révélatrice de leur inadéquation face aux défis et crises que doit surmonter l'Union européenne. C'est pourquoi le pacte de stabilité et de croissance doit être mis au service des mutations économiques et sociales nécessaires à la réussite des transitions climatique et numérique engagées. Dans cette perspective, il est indispensable de dépasser la seule logique du PIB, qui doit être assortie de nouveaux indicateurs de croissance et de richesse, et de réviser notre approche conservatrice et libérale de l'endettement public. Ce dernier est non pas une charge, mais l'une des conditions pour réussir les transitions nécessaires qui sont devant nous. Pour conclure, monsieur le ministre, mes chers collègues, de grands chantiers s'ouvrent devant nous, mais ils supposent au préalable que nous révisions nos outils de coordination économique, dont cet obsolète programme de stabilité. La parole

il n'y a pas si longtemps, nous nous étions habitués à considérer un taux de chômage dépassant les 10 % comme une fatalité. Comble de l'injustice, le taux de chômage des femmes a même parfois dépassé les 12 %. Il n'y a pas si longtemps, nous nous étions résignés. Le secteur secondaire s'effondrait et notre puissance industrielle semblait destinée à n'être plus qu'un lointain souvenir. Il n'y a pas si longtemps, nous pensions qu'une trajectoire de retour à l'équilibre ne pourrait être présentée et qu'il nous serait impossible de repasser en dessous des 3 % de déficit public. Il n'y a pas si longtemps, nous pensions que l'état de nos finances pudiques et la croissance atone nous rendraient impuissants à affronter les crises qui pourraient nous frapper. Et pourtant Pourtant, mes chers collègues, le chômage continue de baisser comme jamais auparavant. Pourtant, l'emploi industriel repart et connaît un regain de dynamisme, grâce au plan de relance et aux réformes fiscales et réglementaires entamées depuis 2017. Pourtant, nous avions réussi à faire repasser le déficit public en dessous des 3 % pour la première fois depuis le début des années 2000, avant, bien entendu, qu'une crise mondiale d'une ampleur sans précédent ne vienne bouleverser nos efforts et ceux du Gouvernement. Pourtant, nous avons su faire face à la crise mondiale la plus grave depuis la dernière guerre mondiale, main dans la main avec nos partenaires européens, grâce à un plan de relance inédit, qui a non seulement sauvé notre économie du désastre et le pouvoir d'achat des Français, lequel a même progressé sur la période, mais également remis notre industrie sur les rails de la compétitivité et permis de préparer l'avenir. Mais la question que j'entends monter du côté droit de l'hémicycle, c'est : pouvons-nous sacrifier au présent notre avenir et celui de nos enfants ? côté gauche, j'entends dire au contraire que nous n'en faisons jamais assez et qu'il ne faut pas laisser la rigueur imposer ses contraintes. Aux uns comme aux autres, je répondrai que la trajectoire proposée par le Gouvernement porte une vision pour la France qui répond à la double exigence qui vous anime, en dépit de nos désaccords. Elle répondra aux inquiétudes en préservant le soutien nécessaire de l'État dans bon nombre de domaines, tout en présentant une normalisation de nos finances publiques qui permette de préserver les générations à venir. Il tiendra à notre vigilance de parlementaires que nous respections cet engagement. Nous comptons sur vous tous, mes chers collègues, comme vous pouvez compter sur nous. Même tardif, ce débat sur le programme de stabilité est toujours un moment de clarté, qui nous permet de nous positionner sur ces questions essentielles et sur la direction que nous prendrons. Mais ce débat redoublera d'importance au moment de l'examen du projet de loi de programmation des finances publiques. Ce sera pour nous, parlementaires, le véritable moment de nous saisir de ce sujet. Le groupe RDPI sera au rendez-vous ! En attendant, nous continuons d'agir dans cette direction pour soutenir l'emploi et l'activité économique, tout en faisant face aux impondérables. Nous avons voté hier l'augmentation du plafond des heures supplémentaires défiscalisées. Encourager l'emploi et la croissance, rétablir nos finances publiques, soutenir les plus fragiles : telle est la volonté qui nous anime depuis 2017 et c'est l'équation délicate que nous aurons à résoudre au cours des années qui viennent.

C'est une réalité à laquelle il semble difficile de s'opposer, bien qu'on en comprenne facilement les causes. Mais là n'est pas l'essentiel, et ce pour au moins deux raisons. La première, c'est que le calendrier électoral a percuté la procédure européenne. Certes, le Gouvernement a bénéficié d'une certaine forme de stabilité, notamment à Bercy, ce qui aurait pu lui permettre d'être dans les temps, mais on aurait tort d'ignorer ce qui s'est passé depuis le mois d'avril dernier. La majorité présidentielle est désormais prise en tenaille entre deux mâchoires populistes, l'une à l'extrême droite, l'autre à l'extrême gauche. Cette configuration commande la prudence. La seconde raison, mes chers collègues, c'est qu'au fond nous connaissions déjà la teneur de ce programme de stabilité. C'est une question de mathématiques : deux points ne peuvent être reliés que par une seule droite. Autrement dit, connaissant la situation actuelle de nos comptes, soit le point de départ, et le point d'arrivée fixé par le Gouvernement- un déficit inférieur à 3 % du PIB en 2027 -, il n'y a guère qu'une seule trajectoire À mes yeux, les débats se cristallisent autour d'un seul mot : la dette. Mais ce mot peut être qualifié par plusieurs épithètes. Je vous en propose quatre : il y a notre dette publique,

non pas simplement la gestion actuelle des comptes, mais aussi, et pour beaucoup, la gestion passée. C'est aussi celui qui nous annonce la quantité d'efforts à fournir dans le futur, que ce soit par la réduction des dépenses ou par la hausse des impôts. Car il faudra bien ramener les dépenses en deçà des recettes, si nous voulons éviter la banqueroute. C'est là non pas une obsession « austéritaire », mais une question de bon sens. L'histoire a montré que les pays qui ne tiennent pas leurs comptes sont rarement ceux qui financent les politiques sociales ou environnementales les plus ambitieuses. En effet ! Le problème n'est pas nouveau, tant s'en faut. Sur ce point, le rapporteur général a raison de nous rappeler, avec une constance irréprochable, la comparaison avec l'Allemagne : plus de quarante points de PIB séparent nos taux d'endettement. Ce décrochage s'explique notamment par une succession d'erreurs politiques et stratégiques passées. Par une Par une funeste inspiration, la France a décidé de sacrifier son industrie sur l'autel des services. Elle a laissé filer ses usines à l'étranger et, avec elles, les emplois qualifiés qu'elles offraient. Résultat : notre balance commerciale, comme notre solde budgétaire, est devenue structurellement déficitaire. Nous avons réuni les conditions d'un endettement fatidique. Avec la pandémie, notre dette publique a explosé. Le « quoi qu'il en coûte », choix tactique rationnel en période de taux bas, risque aujourd'hui de créer un précédent. Il faut vite tourner la page. Il faut, bien sûr, réduire les mesures de soutien temporaire, mais aussi s'attaquer au déficit structurel. Or, à cet égard, monsieur le ministre, je suis au regret de constater que la trajectoire présentée dans le programme de stabilité n'a rien de rassurant. Si le déficit public doit être ramené sous la barre des 3 % du PIB d'ici à 2027, le taux d'endettement, lui, se stabiliserait autour de 113 % du PIB. Il est peu probable que la réalité soit finalement plus favorable que ce qui est prévu dans le programme. Mais cet indicateur, qui sert bien souvent de boussole pour le pilotage des finances publiques, masque deux autres types d'endettement, qui n'apparaissent pas dans le ratio de la dette publique. À la faveur de la crise sanitaire, si l'on peut parler ainsi, et grâce à l'engagement de la France, l'Union européenne s'est, pour la première fois, endettée propre. Cet endettement supra-étatique constitue une avancée majeure pour la construction européenne. Or le Premier Président de la Cour des comptes l'a affirmé devant la commission des finances : le remboursement des sommes versées à notre pays dans ce cadre, qui s'élèvent à 75 milliards d'euros, n'entre pas dans le calcul du ratio de dette publique. Autrement dit, notre dette publique nationale serait encore plus élevée, si nous y intégrions tous les crédits avec lesquels nous avons financé notre plan de relance. il est une autre dette qui n'apparaît pas dans nos comptes publics, et qui a de quoi nous inquiéter. C'est la dette privée, qui concerne à la fois les entreprises et les ménages. Elle avoisine les 150 % du PIB, bien au-delà de la dette publique- c'est colossal En la matière, la France a le taux d'endettement privé le plus élevé des grands pays européens. Le diagnostic est évident : nous sommes plus proches de la Grèce que de l'Allemagne, bien malheureusement. Ce ratio d'endettement privé a ses fondements. Les dispositifs d'urgence mis en oeuvre pendant la crise, ainsi que le contexte de taux négatifs ont encouragé les entreprises à s'endetter massivement pour recruter et investir. Les effets positifs sont donc nombreux. Mais le risque existe que nous ayons massivement financé des entreprises, notamment dans les secteurs des nouvelles technologies, dont les valorisations ont été artificiellement gonflées. Pour parachever ce panorama peu réjouissant, j'évoquerai la dernière facette de notre endettement, la dette climatique. C'est la plus grande urgence, celle qui menace non seulement notre pays, mais la planète entière. Cette dette n'apparaît pas plus dans nos comptes, mais elle ravage nos forêts et tarit nos ressources, en eau notamment. Or, monsieur le ministre, mes chers collègues, un pays ravagé par les flammes et en stress hydrique n'est pas gouvernable. Ce défi suppose donc des investissements massifs, dans un contexte très contraint. L'immense défi de la transition écologique nous impose de changer non pas de logiciel, mais de système d'exploitation pour

réaliser des investissements ambitieux au profit de la transition écologique et des infrastructures locales. Le second levier, plus structurant, mais moins immédiat, c'est une meilleure valorisation des externalités positives et négatives pour mieux orienter les décisions des acteurs économiques, sous la contrainte du changement climatique.

n'était utile qu'une fois abattu. Cela n'est absolument pas satisfaisant. Quand la forêt brûle, cela ne constitue pas seulement un manque à gagner, c'est un atout en moins pour la transition écologique. Je vous proposerai prochainement un dispositif pour prendre en compte les externalités positives de la forêt- puits de carbone, agent de la biodiversité et filtre à eau -et engager ainsi le changement de mode de pensée que j'appelle de mes voeux. En conclusion, monsieur le

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voilà réunis au coeur de l'été pour discuter d'un document stratégique qui va engager la responsabilité du Gouvernement sur sa gestion des finances publiques à moyen terme.

la croissance potentielle est un paramètre déterminant pour la programmation des finances publiques. En effet, elle constitue la meilleure prévision de la croissance du PIB à moyen terme. Mais pour être crédible, l'hypothèse de croissance potentielle doit correspondre à un régime de croissance équilibré.

Les éléments d'analyse rassemblés par un membre du secrétariat permanent du Haut Conseil des finances publiques laissent d'ailleurs penser que, dans les cinq années qui viennent, la croissance potentielle de l'économie française sera plutôt proche de 1 %, ou légèrement inférieure ou supérieure à ce niveau selon le degré de mise en oeuvre de la réforme des retraites. Or le doute est permis sur cette réforme, puisque le président candidat a rétropédalé dès l'entre-deux-tours ... Et le rendement de l'allongement de la durée de cotisation n'est pas le même que celui du report de l'âge de départ. Notre absence de courage aujourd'hui aura des conséquences significatives pour nos enfants et nos petits-enfants. En effet, les projections du Conseil d'orientation des retraites (COR) indiquent que le taux de remplacement, et donc le niveau de vie des retraités, passerait de 102,8 % du niveau de vie des actifs en 2020 à 82,5 % en 2070.

Permettez-nous d'être inquiets, car le plan de stabilité repose uniquement sur ce qui ne dépend pas complètement de l'action du Gouvernement- la baisse de l'inflation, le maintien de la croissance -plutôt que sur la maîtrise des dépenses publiques, sur laquelle il a complètement la main.

l'élargissement de l'apprentissage aux lycées professionnels, par exemple. Certes, le succès de cette politique ne m'a pas échappé : le taux d'emploi des jeunes s'est considérablement amélioré, mais au détriment de la productivité de notre économie et avec un coût important

la mise en place d'un service public de la petite enfance est bien une nécessité. Comme l'indique le programme de stabilité, les prestations familiales ont considérablement diminué, de 3,7 %, du fait de la faible natalité de ces dernières années.

environnemental (CESE) de mars 2022, il n'existe pas de places d'accueil formel pour 40 % des enfants de moins de trois ans. Nous assistons à une érosion de l'attractivité de ces métiers, un mouvement si fort qu'il conduit un nombre important de collectivités locales à « geler » des berceaux. Et ce n'est pas l'ordonnance du 19 mai 2021 sur les services aux familles ou le comité de filière que vous avez institué en 2021 qui apportent une réponse : il ne s'agit que d'un début de réponse. D'ailleurs, l'avis du CESE de mars 2022 plaide pour la mise en place d'un droit opposable à la garde du jeune enfant, comme ce qui a été institué par l'Allemagne en 2004.

euros. Au-delà de quelques exemples précis, que l'on peut compter sur les doigts d'une main, les propos relatifs à la maîtrise de la dépense sont très généraux dans ce document. Il y est question de « renforcement de la qualité des dépenses

Dans les perspectives économiques publiées en juillet 2022, l'OCDE appelle le Gouvernement à mettre en place une stratégie ciblée d'assainissement budgétaire à moyen terme, en fixant des priorités claires pour sauvegarder la viabilité des finances publiques et l'efficience de la dépense publique dans un contexte de hausse du service de la dette. Permettez-moi de vous dire que nous n'y sommes pas encore ! Dans votre stratégie, j'ai du mal à voir quel sera l'effort réellement demandé aux collectivités territoriales. Le programme de stabilité évoque une concertation, comme le ministre Béchu le disait lui-même il n'y a pas si longtemps dans cet hémicycle.

vous laissez simplement les collectivités codéterminer les modalités de modération de leurs dépenses, et l'effort demandé est beaucoup plus important que celui qui avait été demandé par les contrats de Cahors.

sauf à augmenter les impôts locaux, ce qu'elles vont avoir de moins en moins la capacité de faire avec la suppression de la taxe d'habitation et, demain, de la CVAE. Je ne dis pas que nous sommes défavorables à la politique de réindustrialisation. Au contraire, nous pensons qu'il est nécessaire de réduire notre différentiel de compétitivité avec l'Allemagne. Mais nous pensons aussi qu'il est nécessaire de laisser de la liberté aux collectivités territoriales dans la gestion de leurs recettes et de récompenser leurs actions d'attractivité. Notre pays va continuer de diverger avec les autres pays de la zone euro. L'analyse des programmes de stabilité des huit principaux pays de la zone euro menée par la Cour des comptes dans son dernier rapport sur l'état des finances publiques relève que la France serait, en 2025, l'un des rares pays qui n'aurait pas commencé à réduire la dette héritée de la crise sanitaire. L'Italie, l'Espagne prévoient de réduire leur endettement de 10 points de PIB sur la même période. Cette divergence vient du fait que la France aurait le déficit structurel le plus élevé des huit pays étudiés. À l'automne, vous pourrez compter sur nous, et vous nous trouverez pour défendre une mesure simple et concrète pour redresser les comptes publics : la mise en place d'une règle d'or.

il n'est pas besoin de plus de temps pour constater le manque de fiabilité et l'insincérité des hypothèses économiques, largement optimistes et surestimées, qui le sous-tendent. piochez dans la fourchette haute des prévisions, certainement parce que celles de la Banque de France ou des conjoncturistes, plus réalistes, étaient trop embarrassantes. L'effet combiné de ces évaluations en trompe-l'oeil est de surestimer la santé économique du pays et, hélas, de sous-estimer les difficultés des ménages dans les années à venir.

Il n'y a pas de surprises dans ce texte, tant il est pétri d'orientations néolibérales et de mesures antisociales basées sur des réformes structurelles, telles que l'aménagement des retraites et de l'assurance chômage, et prises pour faire des économies, alors même que l'effet que vous en espérez est loin d'être certain. Faute d'agir sur les recettes, comme nous le préconisons, et d'appliquer une fiscalité plus exigeante sur les hauts revenus et les profits, vous continuerez à faire peser sur les classes moyennes et populaires les frais de cette politique, puisque les revenus de transfert et l'accès aux services publics diminueront, ce qui provoquera, à terme, un creusement des inégalités. Ne nous leurrons pas, contrairement à ce qui a été affirmé, les collectivités ne seront pas épargnées par cette politique austère, alors que beaucoup d'entre elles sont déjà exsangues.

Les préconisations de votre programme de stabilité feront donc inévitablement pâtir la qualité du service public, auquel vous allez porter un coup fatal, alors qu'il garantit le dernier lien avec certains de nos concitoyens les plus précaires. précaires. Surtout, l'austérité qui sous-tend ce programme de stabilité n'est pas compatible avec l'impératif de conversion écologique. En autorisant des hausses ciblées sur les secteurs prioritaires que sont les armées, l'intérieur, la recherche, la justice et l'aide publique au développement, ce document le secteur de l'écologie, qui a pourtant cruellement besoin de financements publics. Malgré votre obstination à en faire un détail de l'histoire, il n'est pas acceptable, il est même dangereux de continuer à vous engluer dans l'inaction climatique, en ne prévoyant pas de mesures à la hauteur d'un des plus grands défis que nous ayons à affronter. La programmation que vous nous présentez est climaticide. Il fallait un changement de paradigme clair. Vous en êtes incapables, comme les débats que nous avons eus il y a peu sur le PLFR l'ont, encore une fois, démontré. Vous auriez pourtant pu financer ces dépenses indispensables à notre avenir par les mesures fiscales justes que nous vous proposions, et que d'autres proposaient également : un ISF climatique ou une contribution des superprofits des multinationales. Mes chers collègues, ce que ce document ne dit pas est plus important que ce qu'il dit : l'austérité est devant nous, alors que les besoins sociaux et environnementaux sont criants. Nous ne pouvons avec sincérité donner caution à ce programme insincère. Monsieur le ministre, vous vous entêtez dans un système idéologique délétère, sans tirer les leçons du passé et en voulant obstinément respecter les impératifs budgétaires de Maastricht. Pourtant, le seuil de 3 %, dépourvu de fondement économique, avait été jugé dépassé par le Président de la République lui-même.

monsieur le ministre, d'être lucide sur l'incompatibilité structurelle entre les besoins d'investissement public immédiats et ambitieux que la transition écologique nous impose et les règles budgétaires européennes, qui entravent nos capacités de dépenses publiques. Mener deux combats de manière simultanée condamne irrémédiablement à échouer dans les deux. Il est grand temps d'avoir le courage de mettre en place une politique de soutenabilité budgétaire fondée sur un principe de soutenabilité économique et environnementale, et non pas seulement sur des critères comptables. Vous m'avez donc compris, mes chers collègues, nous refusons un programme de stabilité qui est obsolète avant même d'avoir été mis en oeuvre, un programme dont l'optimisme est si farouche qu'il confine à la malhonnêteté et amorce des mesures dévastatrices face aux enjeux de taille qui se profilent.

cette clarification aurait stimulé le débat critique et la démocratie. Les électeurs auraient pu constater le peu d'égard d'Emmanuel Macron pour la question sociale. Le verdict est tombé fin juillet, trois mois après le délai prévu par les textes, au grand dam du Parlement et du Haut Conseil pour les finances publiques. Ce programme de stabilité est déjà dans la boîte aux lettres de la Commission européenne. Dès lors, impossible de l'infléchir. Le débat est clos. Nous ne sommes plus à un retard près, mais, croyez-moi, la démocratie parlementaire saura s'en souvenir. Le programme de stabilité, dans le jargon, est censé décrire les moyens mis en oeuvre pour respecter la contrainte des règles budgétaires européennes et maintenir le déficit en deçà de 3 % du PIB. D'un point de vue politique, c'est un document annuel, dans lequel le Gouvernement prête allégeance à l'Union européenne, en lui donnant des gages de libéralisme pour attester d'un prétendu sérieux budgétaire. La perspective n'est pas réjouissante, tant la crise sanitaire et la crise économique à dominante inflationniste ont engendré des dépenses pour partie incontournables, mais jamais financées.

Cet héritage nous conduira à l'impasse, rendant les objectifs économiques, sociaux et écologiques inatteignables. Comment ne pas voir au moins un paradoxe, et plus certainement un contresens,

Ces décisions nous rendent tributaires du niveau général des prix de la zone euro et nous placent sous le joug de nos créanciers, qui ne vont pas manquer de réclamer leur dû ! Il nous faudra faire baisser l'inflation par des politiques de rigueur pour éviter que, comme cette année, 17 milliards d'euros supplémentaires ne soient versés aux spéculateurs sur les titres du Trésor. Le Gouvernement évoque un plan : il suffirait de soutenir la croissance et de réduire les dépenses pour compenser les pertes de recettes. Mais le Haut Conseil des finances publiques, tout comme les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est particulièrement sceptique sur les prévisions de croissance.

C'est une aberration fondamentale : les privés d'emploi seraient responsables de leur sort ; le patronat, lui, serait exempt de toute injonction. Ces réformes, nous les combattrons les unes après les autres, mais avec des propositions alternatives. La réforme de l'assurance chômage s'est abattue sur plusieurs millions de travailleurs. Un seul effet : plus d'ouverture ou de rechargement de droits pour les périodes en emploi de moins de six mois. Ces gens travailleraient, mais pas assez ! Regardez la réalité de ce que vous appelez le marché de l'emploi : en 2021, près de 15 millions de contrats de moins d'un mois ont été signés,

Monsieur le ministre, mes chers collègues, comptez sur notre mobilisation : il n'y aura pas d'acte II de la réforme de l'assurance chômage, car c'est l'un des piliers de notre modèle social. La réforme des retraites est une réforme injuste, brutale, de l'avis de toutes les organisations syndicales. Heureusement, elle n'a pas encore eu Loin de la réforme systémique, abandonnée après un mouvement social d'ampleur et grâce à une majorité de rejet, une réforme paramétrique avec un report de l'âge de départ à la retraite à 65 ans est réapparue dans la campagne présidentielle. Il faudrait travailler plus longtemps pour financer les cotisations d'un nombre de retraités plus important.

Les faire travailler plus longtemps va réduire les versements de l'assurance vieillesse au détriment de l'assurance chômage et plus l'âge reculera, plus le chômage augmentera. La belle affaire

Bref, mes chers collègues, la réforme des retraites n'a pas vocation à combler le déficit des retraites, mais à financer d'autres dépenses sociales. Bruxelles et les marchés financiers le demandent et le Gouvernement s'en réjouit.

Remettons les gens au travail, quoi qu'il leur en coûte, voilà votre doctrine ... Le Haut Conseil des finances publiques vous le dit : « L'impact de ces réformes paraît nettement surestimé, puisqu'il est présumé se manifester dès 2023, alors que toutes les réformes comparables entreprises dans le passé ont non seulement nécessité du temps pour leur formalisation et leur mise en oeuvre, mais également pour produire des effets durables sur la population effectivement en emploi. » Alors, monsieur le ministre, nous sommes là parce que satisfaire Bruxelles et les marchés financiers sur le dos des travailleurs, sur le dos des Français, est une orientation politique aux antipodes de nos valeurs et de nos aspirations.

Ce retard est d'autant plus regrettable que notre pays assurait alors la présidence du conseil de l'Union européenne et qu'il eût été intéressant que ce programme nous soit présenté au moment du débat national des élections législatives. Ce retard traduit aussi un certain manque de respect du travail du Parlement et de sa mission essentielle d'évaluation et de contrôle. Nous devons examiner à la hâte ce document, alors qu'il est essentiel puisqu'il dessine la trajectoire des finances publiques pour toute la durée du nouveau quinquennat.

comme il y a cinq ans, vous prévoyez un taux qui doublerait sur la durée de la mandature, passant de 1,25 % à 2,50 %. Vous partez d'une prévision supérieure à celle de la Commission européenne, qui mise quant à elle sur un taux plus raisonnable de 1 %. Vous pariez même sur une accélération de la croissance du PIB, qui atteindrait 1,8 % en 2025. Celle-ci résulterait des réformes engagées, notamment celles des retraites et de l'assurance chômage, dont nous savons qu'elles ne produiront tous leurs effets qu'à moyen terme. Nous savons également que le calendrier n'est pas fixé ; nous ne savons pas quand ces mesures s'appliqueront ni combien elles rapporteront. Comment pourrions-nous être en mesure d'en évaluer l'impact sur les finances publiques ? Enfin, un rapide coup d'oeil sur l'évolution du ratio entre les prélèvements obligatoires et le PIB montre que la pression fiscale ne diminuera pas, contrairement à ce qu'on laisse croire aux contribuables français. français. Le Gouvernement annonce baisser les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les impôts et les cotisations sociales. Or, si l'on en croit le projet de programme de stabilité pour les années 2022 à 2027, le taux de prélèvements obligatoires resterait pratiquement stable jusqu'à la fin du quinquennat. En réalité, les baisses concédées et affichées comme telles dans le discours politique du Gouvernement correspondent à des rétrocessions partielles de recettes fiscales, lesquelles augmentent spontanément du fait de la conjoncture économique. Mais ces baisses ne correspondent aucunement à des baisses structurelles d'imposition. Et pour se permettre de telles baisses, encore faudrait-il être en mesure de diminuer les dépenses publiques, sauf à rejeter avec inconscience le fardeau des déficits et de la dette publique sur les épaules des générations futures. Nous avons aujourd'hui un ratio de dépenses publiques sur PIB de 57,3 %, ce qui est le reflet d'un État qui dépense trop et surtout qui dépense mal,

Nous pouvons y lire qu'une réduction des dépenses publiques de l'ordre de 8 milliards d'euros par an est attendue à partir de 2024. À quoi correspondent ces milliards ? D'où viendront, concrètement, ces économies ? Au Sénat, nous sommes particulièrement vigilants sur la trajectoire proposée pour les collectivités locales. mentionne une réduction des dépenses de fonctionnement de l'ordre de 0,5 % en volume, sans plus de précisions. Or Emmanuel Macron, alors président candidat, a annoncé faire peser sur les seules collectivités territoriales un effort de plus de 10 milliards d'euros sur cinq ans.

Monsieur le ministre, quels seront les objectifs fixés aux collectivités territoriales ? Les contrats de Cahors, cette contribution des collectivités au redressement des comptes publics, vont-ils être ressuscités ? Les élus locaux, dont nous sommes au sein de la Haute Assemblée les relais, y voir beaucoup plus clair. Le groupe Union Centriste et mes collègues ici présents Sylvie Vermeillet et Michel Canévet ont eu l'occasion d'insister sur ce point tout au long de la discussion du PLFR. Nous sommes tout particulièrement inquiets par l'emballement de notre endettement public.

Il y a urgence à ce que nous fixions collectivement un cap de redressement de nos comptes publics afin d'éviter que l'État et, finalement, les Français ne se retrouvent en situation de ruine. La parole

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, proposer chaque année un programme de stabilité, tenir les promesses qu'il contient ou même s'en approcher, est-ce un exercice vain ? La fin de la pandémie annonçait des jours meilleurs sur le plan économique, jusqu'à ce que la guerre en Ukraine vienne repousser cet espoir. Comment prévoir de l'économiquement stable dans un environnement géopolitique instable ? L'équation est difficile ... À la lecture du programme de stabilité 2021-2027 2021-2027 transmis l'année dernière à Bruxelles, il était question d'un rebond de l'activité économique de 4 % en 2022, puis de 2,3 % en 2023. ministre, nous devrions nous contenter d'une croissance de 2,5 % cette année et de 1,4 % l'année prochaine. À la fin de l'année 2021, l'évolution de la situation sanitaire demeurait le principal aléa. Mais voilà, nous faisons face aujourd'hui à une crise sévère des prix de l'énergie et des matières premières. Comme on le sait, il en résulte une inflation très forte- près de 5 % -, un niveau de plus en plus difficile à supporter pour nos concitoyens les plus modestes, sans oublier les entreprises, qui doivent brutalement gérer des hausses de coûts de production. Dans ces conditions, quelles sont les nouvelles perspectives pour les années 2022 à 2027 ? grâce à un ajustement structurel de 0,3 point de PIB par an à compter de 2024. Vous comptez aussi contenir la dette à terme. Certains diront que vous péchez par excès d'optimisme. La Cour des comptes a exprimé ses doutes, en effet, sans toutefois remettre en cause votre stratégie à deux jambes : soutien à la croissance et maîtrise des finances publiques. Si la politique du « quoi qu'il en coûte » a été essentielle à la stabilisation de notre économie, il est temps de revenir à une certaine modération, sans toutefois gripper la croissance, en particulier son principal moteur, la demande.

la revalorisation des pensions de retraite et d'invalidité, des prestations familiales, des minima sociaux et des bourses étudiantes, ainsi que la revalorisation du point d'indice de la fonction publique. Il est sûr néanmoins que certaines de ces mesures n'ont pas vocation à durer. Aussi, l'un des principaux enjeux de votre programme de stabilité, vous l'avez clairement affirmé, est l'emploi- plus précisément, le plein emploi.

Toutefois, je m'interroge sur le retour au plein emploi et sur vos hypothèses de productivité : la croissance potentielle ne sera pas forcément la croissance acquise. Sur le volet maîtrise des dépenses publiques, je rappellerai tout d'abord que mon groupe n'est pas composé d'ayatollahs de l'orthodoxie budgétaire. Les politiques d'austérité ne mènent jamais bien loin- nous l'avons constaté après la crise de 2007-2008. À ceux qui les prônent, rappelons que l'Union européenne elle-même s'en écarte désormais assez facilement. Certes, la dette doit redevenir soutenable. C'est une responsabilité que nous avons à l'égard des générations futures, d'une part c'est un enjeu de crédibilité de l'économie française, d'autre part. Il faut apaiser les tensions sur nos obligations souveraines. Le Gouvernement souhaite que les dépenses en volume de l'État ne progressent pas de plus de 0,4 % par an. Pour certains, cet effort n'en est pas un. Il est vrai que, à l'horizon de 2027, la dette restera encore élevée, avec un taux de plus de 112 % du PIB. question : comment faire autrement, alors que beaucoup de nos services publics ont des besoins immenses, qu'il s'agisse de l'éducation, qui n'est pas simplement une dépense de fonctionnement, mais aussi un investissement pour l'avenir, de la santé ou de la police ?

Je n'oublie pas les collectivités locales, qui doivent conserver les moyens de poursuivre leur action. Certaines- on l'a bien vu en temps de crise -constituent un amortisseur social. Les associations d'élus s'inquiètent des nouvelles contraintes que leur impose le programme de stabilité, à savoir une augmentation de leurs dépenses de fonctionnement inférieure de 0,5 % par rapport à leur tendance naturelle, alors que l'inflation pèsera lourdement sur leurs investissements. Monsieur le ministre, au regard d'un équilibre à trouver entre soutien à la croissance et maîtrise des finances publiques, la question des impôts

Certes on ne peut ignorer que la France apparaît au sein de l'Union européenne comme le mauvais élève concernant le poids de ses prélèvements obligatoires. C'est un fait ! Cependant, il est bon de rappeler dans le même temps que les États membres se livrent encore aujourd'hui à une concurrence fiscale intra-européenne dont la France ne sort pas gagnante. Quand nous mettons en place un impôt sur les grandes fortunes, des particuliers s'installent en Belgique. Quand les impôts sur les sociétés sont trop élevés, les entreprises déportent leur siège en Irlande. Par conséquent, la Commission européenne doit s'attaquer plus frontalement au problème du manque de coordination des politiques budgétaires. Cela suppose, comme le groupe du RDSE le rappelle régulièrement dans les débats sur l'Europe, de revoir la règle de la majorité qualifiée pour certaines décisions, en l'occurrence fiscales. Le véto hongrois sur la taxation minimale internationale des entreprises illustre cette nécessité urgente. Les dernières crises ont montré que les solutions passaient de plus en plus par l'Europe et par la solidarité qu'elle est capable de mettre en place au bord de l'abîme. Les prochains mois s'annoncent encore difficiles, en particulier pour certains pays- je pense à l'Italie -et les écarts de taux d'intérêt menacent la cohésion au sein de l'Union. Le programme de stabilité dont nous débattons aujourd'hui est une sorte de boussole demandée par Bruxelles. C'est un engagement européen que chaque État prend dans son coin, au risque que les boussoles n'indiquent pas toutes la même direction. Resserrer les rangs entre les États membres est donc fondamental. La

c'est avec des finances publiques parmi les plus dégradées de la zone euro que nous entamons ce nouveau quinquennat. Nous héritons d'un déficit public plus de deux fois supérieur à celui de 2017 et d'une dette publique qui a progressé de 17 % en cinq ans. La cote d'alerte est atteinte. Nous étions nombreux à le penser ; nous voilà confortés dans notre diagnostic, dont vous contestiez la pertinence il y a quelques mois, Il est donc de notre responsabilité d'aborder ce débat avec lucidité et prudence. Lucidité quant aux effets de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt sur la dette ; l'horizon est non pas à cinq ans, mais plutôt à dix ou quinze Prudence sur les prévisions qui fondent la vision stratégique que vous nous proposez : le Haut Conseil des finances publiques a rappelé leur fragilité. Le cycle inflationniste ne s'éteindra pas l'an prochain, ni même dans quatre ans, tant les raisons structurelles qui le portent sont fortes et cumulatives. Il faudra donc « dépenser bien, dépenser utilement », comme vous l'avez dit, monsieur le ministre.

l'effort demandé aux collectivités sur leurs dépenses de fonctionnement serait de 15 milliards d'euros sur les cinq prochaines années par rapport à l'année 2022. L'encadrement de l'autofinancement et L'encadrement de l'autofinancement et de l'évolution des recettes réduira l'offre de services à la population et constituera un risque pour le pouvoir d'achat, dans un contexte où la consommation des ménages recule. L'encadrement des dépenses de fonctionnement apparaît contradictoire, dans un contexte de relance marqué par le besoin d'investissement et de soutien aux acteurs locaux. En 2021, les soldes d'exécution des collectivités étaient proches de zéro. Il est donc incompréhensible et inconcevable qu'elles continuent à être pénalisées. Encadrer ces dépenses reviendrait à reproduire les erreurs du passé.

qui est même reparti à la hausse, en volume, depuis 2018. Les collectivités se voient imposer depuis trop longtemps la formule « essayer de faire mieux avec moins ». Les efforts ne peuvent pas, de nouveau, reposer sur elles. Dans un contexte marqué par une inflation record, les communes attendent à l'inverse une revalorisation de leurs recettes pour assurer la continuité des services publics locaux essentiels à la population. Une réponse rapide est possible. Nous devrons l'aborder lors de l'examen de la loi de finances. Comme ce fut le cas

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le programme de stabilité 2022-2027 soumis au Parlement dresse la trajectoire et les perspectives pour nos finances publiques à l'horizon de 2027. Il est marqué par les conséquences de la guerre en Ukraine, les tensions inflationnistes, l'impact des mesures du Ségur de la santé et les dispositifs d'urgence liés à la crise sanitaire. Les administrations de sécurité sociale, qui représentent la moitié de la dépense publique, devront participer à la modération des dépenses, au même titre que l'État et les collectivités territoriales, dans un ratio de 0,6 % par an en volume. Les finances sociales ont supporté la crise sanitaire.

La santé demeure la priorité numéro un des Français. Nos urgences, nos hôpitaux, le personnel qui y travaille sont depuis longtemps installés dans une situation critique, devenue insupportable. L'accès aux soins reste compromis dans de nombreux territoires. Face aux dépenses qu'impliquent ces enjeux légitimes et dans le respect d'un budget équilibré, la voie sera étroite pour trouver et financer les solutions attendues. Le défi est grand : faire plus avec autant Monsieur le ministre, au sein du groupe Union Centriste, nous soutenons plusieurs positions complémentaires à la réforme des retraites, système complexe et fragmenté, sollicitée par la Commission européenne.

les Français y sont de leur poche pour 2,7 milliards d'euros, soit 2,6 % du montant des frais de santé. En ce qui concerne ensuite la pertinence des soins, le rapport de Jean-Marie Vanlerenberghe de 2017 souligne qu'une part d'interventions sans valeur ajoutée pour la santé constitue une forme de économiques (OCDE) évalue à peu près à un cinquième des dépenses de santé. Les voies d'économies sont connues. Elles correspondent à des soins inadaptés, tels que des césariennes ou des examens d'imagerie non justifiés, des surprescriptions d'antibiotiques ou encore le recours aux urgences hospitalières inutile ou évitable. Enfin, la troisième voie d'économies est la lutte contre la fraude. Tant notre collègue Nathalie Goulet que de nombreux rapports dénoncent l'existence d'une fraude importante. Nous entendons que les caisses de Sécurité sociale y travaillent. Toutefois, l'étape de la cartographie des risques n'est pas celle du déploiement d'actions correctrices. La méthode est la bonne, mais il faut continuer d'avancer vite, en traitant l'ensemble des champs. (Ondam) a sans nul doute permis de juguler la dette sociale. Toutefois, l'état de notre médecine, tant à l'hôpital qu'en ville, doit nous forcer à interroger la pertinence de cet outil très singulier à la France. Si nous sommes attachés à l'objectif du programme de stabilité, nous ne pouvons ignorer les politiques publiques concernées.

Aussi, le maintien d'un service, d'une unité ou d'un hôpital de proximité ne peut pas être décidé uniquement sous l'angle budgétaire. Au vu de ces éléments, vous avez dressé tout à l'heure, monsieur le ministre, un tableau idyllique de notre pays et de notre situation financière, tout en fustigeant dans le même temps des formations politiques légalement constituées. Or la réalité est tout autre : la dette publique 2 901 milliards d'euros, soit 11,5 % du PIB, la hausse des prix, de 6,1 % en 2021, ne cesse de s'aggraver, le taux de chômage est de 7,3 % et, enfin, la France est championne du monde des prélèvements sociaux obligatoires, à hauteur de 46 %. Voilà la vérité

Le Sénat n'a pas changé de couleur politique, mais l'Assemblée nationale, elle, a sensiblement évolué. Ainsi, le débat que nous avons eu hier à l'Assemblée nationale n'aurait pu avoir lieu si nous avions présenté le programme de stabilité

des retraites, la réforme de l'accompagnement des demandeurs d'emploi ou encore la réforme du lycée professionnel, pour que le succès de l'apprentissage se vérifie aussi dans la voie professionnelle et scolaire.

La réalité est que 0,6 % de croissance en volume sur le quinquennat représente le plus gros effort consenti depuis vingt ans en matière de dépenses publiques. C'est une réalité.

On voit aujourd'hui à quel point la dette nous prive de marges de manoeuvre. Cette année, elle nous coûte 17 milliards d'euros de plus, l'équivalent du double du budget du ministère de la justice ! Si nous continuons à la laisser filer, elle nous privera tellement de marges de manoeuvre que nous n'aurons plus les moyens d'investir pour la transition énergétique et pour la transition écologique.

Face à une inflation exceptionnelle, nos concitoyens attendent des réponses ciblées et immédiates à leurs préoccupations du quotidien : manger, se déplacer, se chauffer, pouvoir concrétiser leurs projets et travailler plus, pour ceux qui le veulent, selon leurs priorités et les possibilités de leur employeur. En examinant ce projet de loi, nous avons veillé à suivre cette boussole, étant entendu que la protection de notre niveau de vie relève de responsabilités partagées : l'État, les collectivités territoriales, que je salue, mais surtout les entreprises et bien sûr les ménages, qui prennent aussi leur part pour faire face à ces augmentations. Même s'il a validé la revalorisation anticipée au 1 juillet de diverses prestations et aides sociales, le Sénat, attentif à l'équilibre financier global des mesures qu'il a adoptées, a tenu à marquer la fin du « quoi qu'il en coûte La commission mixte paritaire, réunie seulement trois jours après l'adoption du projet de loi par le Sénat, est parvenue à établir un texte commun à partir de deux copies assez différentes, il faut bien le Pour la partie relevant de la commission des affaires sociales, le texte de la commission mixte paritaire (CMP) reprend plusieurs apports importants du Sénat sans lesquels le projet de loi n'aurait pas répondu à nos attentes. Tout d'abord, il inclut l'article 1 , que nous avons introduit afin de limiter, de manière pérenne, le surcoût associé aux heures supplémentaires, tout en recentrant ce dispositif sur les petites et moyennes entreprises de moins de 249 salariés. Au travers de ce dispositif, très complémentaire de la réduction d'impôt qui figure dans le projet de loi de finances rectificative, il s'agit bien sûr de rendre effectifs les gains de pouvoir d'achat que les salariés volontaires pourront tirer des heures supplémentaires. La CMP a adopté la mesure de déblocage exceptionnel de l'épargne salariale, qui apportera un soutien immédiat aux salariés dont les revenus sont insuffisants face à la hausse des prix. Elle a également introduit l'accélération de la procédure d'extension des accords salariaux lorsque plusieurs revalorisations du SMIC sont intervenues dans les douze derniers mois.

en particulier la limitation du fractionnement de la prime à un versement par trimestre et l'anticipation du dispositif à la date du 1 juillet 2022. Par ailleurs, la possibilité de cumul entre l'exonération dont bénéficient les jeunes agriculteurs et la réduction du taux de cotisation maladie-maternité, adoptée par le Sénat sur l'initiative de notre collègue Laurent Duplomb, que je salue, a été transformée d'un commun accord en droit d'option pour l'un ou l'autre de ces dispositifs. Les modifications apportées par le Sénat à l'article 3, qui tend à faciliter le développement de l'intéressement, ont été conservées en CMP, en particulier celle qui visent à limiter à quatre mois le délai donné à l'administration pour l'agrément d'un accord de branche d'intéressement, de participation ou instituant un plan d'épargne salariale. La CMP a prévu que ce délai pourra être prorogé une fois, pour une durée maximale de deux mois. Enfin, je me réjouis que l'assouplissement temporaire des règles d'utilisation des titres-restaurant ait été conservé dans la rédaction issue du Sénat. Cette mesure ne doit pas susciter l'inquiétude des professionnels concernés : il me semble que l'équilibre global des aménagements apportés au dispositif du titre-restaurant ne leur porte pas préjudice. Toutefois, j'ai parfaitement saisi l'inquiétude bien plus large du secteur de l'hôtellerie-restauration, sur lequel nous devons porter un regard attentif. Ce texte n'épuise pourtant pas le sujet du pouvoir d'achat. Nous ignorons comment évoluera l'inflation et nous ne savons pas quelles nouvelles mesures seront nécessaires. En outre, nous ne méconnaissons pas la situation singulière des Français les plus fragiles, que ce soit dans les outre-mer ou dans les territoires ruraux. textes devront contenir des mesures plus structurelles en faveur du pouvoir d'achat des Français. Dans l'attente de ces prochains rendez-vous, je vous invite aujourd'hui, au nom de la commission mixte paritaire, à adopter ce projet de loi. La parole est à M.

Monsieur le président, madame la ministre, madame le rapporteur, monsieur le vice-président de la commission des affaires sociales, madame la présidente de la commission des affaires économiques, mes chers collègues,

Je me réjouis que notre commission y ait imprimé sa marque. De manière générale, nous avons souhaité maintenir un équilibre entre la législation d'urgence, d'une part, et la liberté économique et le droit de propriété, d'autre part. De plus, nous avons souhaité combler certains angles morts en matière de protection des consommateurs et de régulation des marchés de l'électricité et du gaz, ainsi que de promotion des solutions de remplacement aux énergies fossiles. C'est fondamental face à la crise inflationniste actuelle.

De plus, nous avons associé les collectivités locales à tous les dispositifs pertinents, parmi lesquels figure l'interruptibilité. Enfin, nous avons circonscrit le champ des méthaniers flottants et complété leur programme d'investissements. Plusieurs apports sénatoriaux ont été pris en compte : tout d'abord, les projets de biogaz bénéficieront de solutions de simplification. En outre, les consommateurs d'électricité et de gaz

Les nouvelles modalités de résiliation des offres groupées, de l'assurance emprunteur et des services de télévision et de vidéo à la demande sont des avancées concrètes. Il en va de même avec la pénalisation des banques, à proportion des retards de remboursement des victimes de fraudes. Bien sûr, ces mesures, techniques et ponctuelles, ne répondent en rien au besoin d'une vision politique et de mesures structurelles.

Nous arrivons au terme de l'examen de ce texte en faveur du pouvoir d'achat des Français, après plus de trois semaines de débats nourris. Je crois que nous pouvons collectivement saluer l'adoption de ce texte qui favorisera le pouvoir d'achat des Français,

ses responsabilités. Je l'ai dit ici même, nous sommes engagés dans une course contre la montre, afin de sécuriser nos approvisionnements en énergie pour l'hiver prochain. Les mesures prévues au titre III du texte donnent à l'État les leviers indispensables pour agir au plus vite.

aux coupures d'énergie pour impayés. Le Parlement apporte une protection supplémentaire aux Français en dehors de la période de trêve hivernale, en instaurant une période incompressible d'au moins un mois avant que la coupure de courant soit effective. Cette période doit être mise à profit pour trouver un accord entre entre le consommateur et le fournisseur. Je salue l'adoption des mesures visant à sécuriser le rehaussement du plafond de l'Arenh de 20 térawattheures. Là encore, un compromis sécurise la protection des entreprises électro-intensives et des collectivités territoriales face aux hausses des prix de l'énergie

Nous avons avancé les revalorisations des prestations sociales prévues au 1 janvier ou au 1 avril prochain. L'ensemble des prestations augmentera de 4 %. Cette revalorisation s'ajoutera à celle de 1,1 % décidée le 1 janvier dernier ou à celle de 1,8 % arrêtée le 1 avril dernier. C'est le cas, entre autres, des minima sociaux, mais également de la prime d'activité. Sur ce sujet, la volonté du Gouvernement est sans ambiguïté : nous n'opposons pas la valeur travail au soutien à nos concitoyens les plus fragiles. Nous avons ainsi proposé, à l'article 3, de favoriser le recours à l'intéressement,

Une instruction confirmera prochainement ces modalités d'application. Ensuite, l'article 4, qui permet d'engager la restructuration des branches professionnelles disposant de minima conventionnels durablement inférieurs au SMIC a été rétabli.

Enfin, les heures supplémentaires bénéficieront d'une nouvelle exonération forfaitaire de cotisations sociales patronales. Cette proposition pérenne s'appliquera aux entreprises de 20 à 250 salariés. Je suis satisfaite qu'un compromis ait pu être trouvé entre les deux chambres sur ce sujet qui allie compétitivité et pouvoir d'achat.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, face à la hausse de l'inflation, une grande partie des Françaises et des Français s'inquiètent de voir leur situation économique se dégrader. Les salariés les plus faibles, les « premiers de corvée », sont et seront frappés de plein fouet. Ce texte censé assurer la protection du pouvoir d'achat constitue un espoir pour eux. Vous disiez vouloir revaloriser le travail. Or tout travail mérite salaire : c'est le contrat social entre l'employeur et le salarié. Les conquêtes sociales et le droit du travail garantissent une juste rémunération qui assure le pouvoir de vivre,

les salaires. Comme nous le redoutions, vous avez ignoré la question salariale dans ce texte sur le pouvoir d'achat. Les revalorisations des prestations familiales, des minima sociaux, de la retraite de base, des APL et du point d'indice des fonctionnaires seront vite rattrapées par l'inflation. la collusion entre le Gouvernement et la droite sénatoriale ne fait aucun doute. Ensemble, vous mettez en oeuvre une politique libérale. Ensemble, vous faites le choix de la prime au détriment des salaires. Ensemble, vous engagez la déconstruction du statut de salarié. La prime Macron, désormais injustement appelée prime de partage de la valeur, n'est versée qu'à la discrétion de l'employeur et par une minorité d'entreprises : seuls 10 % des salariés en ont bénéficié, et son montant moyen n'a jamais dépassé les 550 euros. Ce n'est pas en augmentant le plafond des possibles que vous accroissez la prime ou le nombre de bénéficiaires ; c'est un leurre. Cette prime, désocialisée et défiscalisée, va à l'encontre du modèle social que nous défendons. Elle s'éloigne du principe selon lequel chacun contribue en fonction de ses moyens et bénéficie en fonction de ses besoins. Pas de cotisations, pas de droits associés et des comptes de sécurité sociale dégradés : c'est un affaiblissement de notre protection sociale.

de biogaz. Pourtant, les mesures visant à sécuriser l'approvisionnement énergétique en gaz et en électricité ne ressortissent pas au pouvoir d'achat et témoignent du manque d'ambition et de visibilité de la politique énergétique du Gouvernement. Enfin, le relèvement du plafond de l'Arenh de 20 térawattheures dégradera encore plus la situation financière d'EDF, au bénéfice de ses concurrents, qui réalisent de superprofits sans contribuer à la charge commune. Une grande réforme du marché européen de l'énergie est plus que jamais nécessaire. En matière de logement, les dispositions visant à contenir les hausses de loyers ne seront pas assez efficaces pour les usagers les plus modestes.

Nous regrettons que nos propositions visant à valoriser le travail aient été balayées d'un revers de main et sans considération par le Gouvernement et la majorité sénatoriale. Je pense à la valorisation du travail grâce au SMIC qui serait porté à 1 500 euros, à la grande conférence nationale sur les salaires, à la revalorisation des prestations sociales en fonction de l'inflation,

Avec la complicité de la majorité sénatoriale, ... On n'a rien fait ! ... le Gouvernement ne propose que des mesures de court terme, qui ne suffiront pas à répondre à l'urgence sociale dans notre pays.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire réunie le 1 août dernier est parvenue à un accord sur le projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

Ce texte comporte des avancées nécessaires pour protéger efficacement le pouvoir d'achat des Français. Je pense en premier lieu au triplement de la prime de partage de la valeur, qui permet aux entreprises de verser jusqu'à 3 000 euros par an à leurs salariés et jusqu'à 6 000 euros pour celles qui ont créé des dispositifs d'intéressement.

Je pense également à la baisse des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants et les conjoints collaborateurs, ainsi qu'au plafonnement de la hausse des loyers commerciaux, que nous avons défendu avec d'autres groupes.

trop restrictive. La revalorisation anticipée des retraites, du minimum vieillesse, de l'AAH ou de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) s'inscrit dans l'action que nous menons depuis 2017 en faveur du pouvoir d'achat

du RSA est nécessaire, comme le sont les autres revalorisations prévues. C'est bien la preuve de la solidarité nationale vis-à-vis de nos concitoyens les plus modestes et les plus éloignés de l'emploi.

et de la majorité présidentielle se concentre sur une ambition : faire en sorte que chacun puisse trouver un emploi stable et une protection adéquate, afin de vivre dignement. Je pense également au plafonnement des hausses de loyer pour les particuliers, ainsi qu'à la résiliation facilitée par voie électronique des contrats de consommation et à la lutte contre les pratiques commerciales trompeuses. Je pense enfin

Lorsque les enjeux sont d'une importance cruciale pour la vie des Français, nous devons en effet être capables de nous rassembler, quelles que soient les divergences partisanes qui traversent cet hémicycle.

La parole est à M. Franck Menonville, pour le groupe Les Indépendants

madame la ministre, mes chers collègues, selon l'Insee, le pouvoir d'achat des Français devrait reculer de 1 % en 2022, plombé par une inflation galopante qui a franchi la barre des 6 %. doivent faire face à une hausse croissante des prix de l'énergie. Faut-il rappeler que ces derniers ont augmenté de 70 % depuis novembre 2021 Le projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat prévoit de mobiliser 20 milliards d'euros pour soutenir le budget des Français. Je me félicite que ce texte, très attendu par nos concitoyens, ait fait l'objet d'un compromis en

Nos concitoyens ont également besoin de protection au niveau de leurs contrats de consommation et dans leurs rapports avec les banques. Le projet de loi comporte ainsi plusieurs dispositions qui apportent davantage de souplesse. Je pense notamment au remboursement accéléré des fraudes bancaires, au remboursement automatique des frais en cas d'incidents multiples ou encore à l'exonération d'une partie des frais de résiliation anticipée des contrats mobiles et internet. Notre groupe a d'ailleurs défendu des amendements en ce sens. cela ne saurait suffire. La solution à la crise que nous traversons réside, à mon sens, dans le travail, plus particulièrement dans sa valorisation. Alors que de nombreux emplois sont à pourvoir et que les difficultés de recrutement persistent, nous devons nous assurer que le travail paie dans notre pays. Tel est le véritable levier pour améliorer le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Des changements profonds sont nécessaires. En attendant, je tiens à saluer les mesures concrètes adoptées, qui auront un effet positif pour les ménages français.

Troisièmement, le projet de loi favorise l'intéressement dans les entreprises, puisqu'il en assouplit les conditions de mise en place dans les structures de moins de 50 salariés. Le Sénat a également introduit un dispositif de déblocage anticipé de l'épargne salariale jusqu'au 31 décembre 2022.

Dans cette enceinte, nous considérons que la santé financière de nos collectivités territoriales est gage de réussite pour chaque citoyen. Nous resterons donc très attentifs à ce que ces dépenses ne pèsent pas sur nos collectivités,

Vous l'aurez compris, mes chers collègues, ce texte est une bonne nouvelle pour les Français. Le groupe Les Indépendants le votera, mais les défis restent immenses et l'avenir incertain : il nous faudra être au rendez-vous dans les prochains mois. La

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous nous retrouvons cette après-midi pour entériner un accord important, utile et attendu par nos concitoyens. Le texte élaboré par la commission mixte paritaire lundi dernier est le résultat d'un beau travail de nos deux assemblées, capables, lorsqu'elles sont écoutées et respectées, d'enrichir considérablement les projets de l'exécutif. Ni chambre d'enregistrement ni assemblée de blocage, le Sénat a montré tout au long de ces derniers jours sa capacité à trouver des solutions pour soutenir le pouvoir d'achat de nos compatriotes, dans les domaines social, économique et énergétique.

Enfin, nous avons voulu soutenir les ménages les plus modestes, victimes de la crise inflationniste, avec des dispositifs ciblés et rapides à mettre en oeuvre.

Demain, grâce au Sénat, les Français pourront bénéficier d'une prime de partage de la valeur pérennisée, versée au maximum quatre fois par an. Les heures supplémentaires seront encouragées, grâce à une réduction de cotisations Grâce au Sénat, les salariés pourront, d'ici à la fin de l'année, obtenir un déblocage anticipé de leur participation et de leur intéressement dans une limite de 10 000 euros. Il s'agit d'une véritable mesure en faveur du pouvoir d'achat et d'encouragement du travail, dont nous pouvons être fiers. Grâce au Sénat, les ménages en situation de précarité pourront, lorsqu'ils ne sont plus en mesure de payer leurs factures d'électricité, choisir de réduire la puissance plutôt que de subir une coupure sèche de leur alimentation, et ce tout au long de l'année. Grâce à la détermination du Sénat et à la mobilisation de nombreux groupes à l'Assemblée nationale, l'allocation aux adultes handicapés sera enfin déconjugalisée. Mais que de temps perdu ! Je me réjouis à titre personnel de cette avancée majeure, étant engagé depuis longtemps dans ce combat pour plus de justice. Le Sénat a également obtenu des avancées majeures sur le volet énergie du projet de loi qui nous était soumis. Préoccupés par notre sécurité d'approvisionnement en électricité et par les évolutions désastreuses du dispositif de l'Arenh, nous avons obtenu un compromis, bien qu'il soit fragile. En rehaussant le prix de vente de l'électricité nucléaire d'EDF et en gelant le plafond de l'Arenh jusqu'en 2025, nous envoyons un message très clair au Gouvernement : la situation actuelle n'est plus tenable, et il faut vite une réforme. Nous avons soutenu le développement des terminaux méthaniers, notamment au Havre. Nous avons voté pour l'accélération de la stratégie nationale en faveur du biogaz. Nous avons proposé un dispositif innovant d'économies d'énergies rémunérées et volontaires pour les particuliers. Toutes ces mesures sont utiles, mais elles ne remplaceront pas la mise en oeuvre d'une stratégie de long terme, seule capable de nous permettre de rétablir notre souveraineté énergétique. Mes chers collègues, comme vous le constatez, les acquis du Sénat sont nombreux, et j'allais dire inédits, sur un tel texte.

face à la hausse des prix qui frappe durement les Français les plus modestes, une réaction urgente s'imposait. Depuis juillet, l'inflation culmine à 6,1

alors même que, selon la Banque de France, les taux de marge des entreprises n'ont jamais été aussi élevés depuis 1949. La raison en est simple : comme le souligne l', l'augmentation des profits des entreprises alimente celle des prix. des mouvements spéculatifs misant sur la baisse des approvisionnements énergétiques. Pour quels résultats ? Les bénéfices des entreprises explosent, au point que même l'Agence internationale de l'énergie a appelé à taxer les 200 milliards d'euros de surprofits

17 % des entreprises de moins de 10 salariés l'avaient versée, contre 58 % de celles de plus de 1 000 salariés, plus largement distribuée dans les secteurs où les salaires sont déjà plus hauts, cette prime ne permettra pas d'aider les personnes réellement en difficulté, pour qui la hausse des salaires se révèle la solution nécessaire.

Heureusement pour la sécurité sociale, le Gouvernement se pliera enfin à la loi Veil en compensant le manque à gagner ! Néanmoins, le même Gouvernement qui se montre

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, sans surprise, les députés de la majorité gouvernementale et les sénateurs de la majorité sénatoriale sont parvenus à se mettre d'accord en commission mixte paritaire sur une version commune du projet de loi pour la protection du pouvoir d'achat. Nous avions assisté au Sénat à l'annonce des fiançailles entre la droite et le Gouvernement ; nous pouvons maintenant féliciter les heureux mariés qui se sont dit « oui » ! Le panier de la mariée est pourtant amer !

la revalorisation de 1,1 % des retraites de base, alors que l'inflation s'élève à 6 %. En réalité, il ne s'agit là que de mesures de rattrapage partielles de la perte de pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Le Gouvernement préfère encourager le versement de primes temporaires dans les entreprises, plutôt que d'inciter les patrons à augmenter les salaires. Avec ces primes, il donne aux salariés d'une main ce qu'il reprend de l'autre au niveau des pensions de retraite. Au Sénat, la droite a chargé la dot, en votant de nouveaux reculs sociaux et en ajoutant à la liste des mesures de pouvoir d'achat la défiscalisation des heures supplémentaires et la suppression des cotisations sociales des employeurs sur les heures supplémentaires. s'est aggravée. Pour résumer, grâce au Gouvernement, nos concitoyens ne perdront que 2 % de pouvoir d'achat en 2022, tandis que, avec la droite sénatoriale, ils devront travailler davantage pour gagner autant qu'en 2021 Les efforts sont toujours demandés aux salariés. En revanche, les entreprises et nos compatriotes les plus riches, qui ont profité de la crise, ne paieront pas un euro supplémentaire

Le désengagement de l'État au détriment des collectivités territoriales, ça suffit ! À un moment donné, il faut dire stop aux politiques d'austérité et aux logiques libérales mortifères ! Pour notre part, nous pensons qu'une autre politique est possible. Face à l'inflation et aux spéculations des marchés, nous proposons de bloquer temporairement les prix et, pour ne pas pénaliser nos agriculteurs, d'appliquer un coefficient multiplicateur à l'ensemble des produits alimentaires, afin de tenir compte du prix de vente

Pour les retraités, nous proposons d'indexer les pensions sur l'évolution du salaire moyen, de supprimer la hausse de la CSG décidée en 2018 et de porter à 1 041 euros le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Pour

(CICE), qui ampute le budget de l'État de 20 milliards d'euros par an. En conclusion, le Gouvernement et la droite ont profité d'un texte sur le pouvoir d'achat pour remettre en cause les droits sociaux et refuser de mettre à contribution les plus riches en tapant toujours sur nos concitoyens les plus fragiles. Pour toutes ces raisons, le groupe communiste républicain citoyen et écologiste votera contre ce projet

L'enjeu était primordial, puisque nous connaissons actuellement la plus forte inflation depuis 1985. Si nous pouvons nous réjouir de la réaction rapide du Gouvernement, nous devons toutefois souligner que peu de mesures figurant dans ce projet de loi auront des incidences directes sur le pouvoir d'achat des Français. ne nous trompons pas, l'objectif de ce texte était clairement exposé dans son intitulé : il visait à protéger ce pouvoir d'achat, et non à l'améliorer ; certains pourront le regretter, mais personne ne pourra dire que rien n'a été fait. C'est singulièrement l'article 5 qui produira des effets directs, puisqu'il prévoit une réévaluation de 4 % de l'ensemble des prestations, allocations ou aides individuelles, revalorisées annuellement. Le coût estimé de cette opération est de l'ordre de 4,6 milliards d'euros pour la sécurité sociale- je tiens à le préciser -et de 2 milliards d'euros pour l'État et les collectivités territoriales en 2022 et en 2023.

Concernant le champ des affaires économiques et du développement durable, la philosophie du texte est de protéger les Français, notamment en préparant notre pays à l'hiver, afin de limiter la hausse des prix de l'énergie, ou encore en leur permettant de se défaire de contrats aussi facilement qu'ils peuvent les souscrire.

! Pour ce qui concerne notre souveraineté énergétique, les mesures adoptées vont dans le bon sens au regard de l'urgence qui est la nôtre, mais la question de notre indépendance reste entière, et nous devons la régler rapidement.

à l'issue de ce marathon législatif estival, je ne puis que me réjouir, à mon tour, de l'accord trouvé lundi soir en commission mixte paritaire sur ce projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Comme toujours, les débats au Sénat ont été riches et de bonne tenue, malgré des délais de transmission très courts, et même trop courts, madame la ministre. Le groupe RDSE a apporté sa pierre à l'édifice, avec l'adoption de mon amendement visant à limiter à 3,5 % la variation de l'indice des loyers commerciaux (ILC).

le vote conforme sur la déconjugalisation de l'AAH, que notre groupe soutenait depuis longtemps, ou encore le déblocage de l'épargne salariale. Un compromis a été trouvé à l'article 2, afin de permettre aux jeunes agriculteurs- vous savez combien cette filière m'est chère -d'exercer un droit d'option

Je salue, en outre, les dispositions renforçant la protection des consommateurs face aux pratiques commerciales abusives et aux coûts fixes suscités par la souscription de certains contrats d'abonnement avec engagement. Elles s'inscrivent dans la continuité des initiatives parlementaires prises ces dernières années concernant la lutte contre le démarchage abusif. Enfin, le projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat comporte tout un volet de dispositions relatives à la protection de notre souveraineté énergétique, sur le détail desquelles le temps qui m'est imparti dans cette discussion ne me permet pas de revenir. Retenons que la France et les Français seront mieux armés pour affronter les tensions s'agissant de l'approvisionnement énergétique, en particulier l'hiver prochain. prochain. Ces mesures prises dans l'urgence ne sauraient toutefois nous dispenser d'une politique énergétique de long terme, soucieuse de garantir à la fois des prix raisonnables aux usagers et un approvisionnement sécurisé et plus en adéquation avec les objectifs de lutte contre le changement climatique.

Je pense aussi à mon amendement visant à un meilleur fléchage de l'allocation de rentrée scolaire, notamment en direction des coopératives scolaires, malheureusement déclaré irrecevable, comme de nombreux autres amendements émanant de tous les groupes. Plusieurs d'entre nous souhaitaient également une augmentation du salaire net des personnes les plus précaires qui travaillent. Cependant, malgré ces réserves, les membres du groupe RDSE voteront pour l'adoption des conclusions de la commission mixte paritaire. Conformément

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.